Questions orales. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 119 de monsieur Didier Marie, au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la parole est à monsieur Didier Marie. Merci madame la présidente, monsieur le ministre je voudrais appeler votre attention ce matin sur la question du respect des droits humains par les multinationales et la nécessité d'une réglementation internationale européenne contraignante en la matière, nous nous souvenons tous du drame du Rana Plaza en 2013 qui avait provoqué la mort d'un millier de personnes, hommes, femmes, enfants, ouvriers de l'industrie textile, travaillant pour des marques de vêtements international dont une partie était française chaque jour dans le monde des drames se produisent qui, sans avoir l'ampleur malheureuse et la portée médiatique du Rana Plaza sont, pour chacune, pour chacun d'entre eux, une catastrophe humaine ou environnementale du 23 au 27 octobre dernier un groupe de travail de l'ONU s'est réuni à Genève pour la 3ème fois en vue de l'élaboration d'un instrument juridiquement contraignant sur les entreprises multinationales et des droits de l'homme, les négociations ont confirmé la future rédaction d'untel, traité international, celui-ci contribuerait à résorber la asymétrie endroits entre l'employeur et le salarié il viserait par le principe de responsabilité des entreprises à lutter contre les esclavages modernes et à prévenir les écosystèmes à côté d'autres instruments présents et à venir, comme la lutte contre la corruption et les paradis fiscaux, ce traité serait une belle étape vers un nouvel âge de la mondialisation, ni fermeture ni ultra-libéralisme mais une 3ème voie qui place l'humain au centre du développement, plus de 900 organisations de la société civile soutiennent ce processus débuté en 2014, de nombreuses entreprises, notamment européennes, déjà exemplaire ont saisi le bénéfice d'une compétition loyale comme alternative au dumping social et environnemental et nous sommes 245 parlementaires français de tous horizons politiques avoir appelé le 25 octobre dernier le président de la République à faire bouger l'Europe sur ce dossier alors que la loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères et de noces d'or, votée par le Parlement au printemps 2017, pionnière en la matière, a une place importante dans les discussions, a lieu à l'ONU, et alors que vous avez annoncé à l'Assemblée nationale le 17 octobre dernier que la France sera très déterminé à faire en sorte que cette proposition de traiter soit activé et puisse retenir l'attention désigne Nations-Unies, pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, quel est l'engagement de la France, qui doit être sans réserve au rendez-vous de ce processus historique pour la protection des droits humains fondamentaux quelles initiatives ont été prises par le gouvernement et quelles sont celles à venir pour enfin faire aboutir ces négociations, je vous remercie. Merci monsieur Marie, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires s'étrangère. Merci madame la présidente, monsieur sénateur, vous avez raison et je crois que c'est partagé sur l'ensemble de ces bancs, nul ne peut plus continuer à ignorer les violations des droits de l'homme qui peuvent résulter de l'activité directement directe de certaines entreprises, c'est particulièrement vrai dans dans certains domaines de l'extraction mais vous évoquiez un drame qui avait trait à l'industrie notamment textiles et donc c'est vrai que la France et grâce d'ailleurs au Parlement, a pris des initiatives, j'ai en tête cette proposition de loi qui est devenu loi à l'initiative notamment de Dominique Potier si, si ma mémoire est bonne et qui a permis de commencer à traiter ce sujet-là dans un niveau national après effectivement il y a des enceintes internationales, vous l'avez signalé qui qui ont été mandatés se sont réunis, le groupe de travail intergouvernemental que vous évoquez à travailler, fin octobre, la France d'ailleurs insisté pour que, contrairement à ce qui était prévu dans le projet soumis l'ensemble des entreprises soient prises en compte, pas seulement les entreprises transnationales, en fait, on peut avoir une vision encore plus large, d'autant qu'il y a pas vraiment de définition juridique de cette notion d'entreprises transnationales alors malheureusement, il y a pu avoir de de de consensus ou ou d'accord à l'occasion de cette session d'une part parce que le document préparatoire équatorien qui mis sur la table, a été remis, un peu tardivement et que le contenu était malheureusement trop ambitieux pour qu'on arrive à faire converger la la communauté internationale, donc nous attendons impatiemment la tenue d'une d'une 4ème session pour que les discussions se se poursuivent et qu'on puisse enfin aboutir en tous les cas, la France elle, dès le 26 avril dernier poursuit avec un plan national d'action pour la mise en oeuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux droits de l'homme et aux entreprises et qui s'applique notamment aux droits des salariés et puis naturellement nous sommes très engagés pour la mise en oeuvre principes directeurs de l'OCDE à l'attention aux entreprises multinationales pour qu'elles adoptent un comportement responsable et éthique donc la France soit liaisons assuré Monsieur le de sénateurs, elle est déterminée à poursuivre ses efforts au plan national et international pour porter ce sujet, d'autant que vous évoquiez une 3ème voie et c'est vrai que nous sommes tous un peu sensible à ce qui était la philosophie long bourgeois à la base du solidarisme et qui pose l'humain au centre de tout, donc je crois que c'est un moteur d'ailleurs de de l'action de ce gouvernement et si pour l'instant, les choses n'ont pas encore débouché au plan international, nous continuons à mettre la pression pour avancer. avancer. Le ministre, monsieur Didier Marie, pour une réponse à Monsieur le Ministre. Oui, je voudrais remercier monsieur le ministre, de sa réponse et dire que les efforts que notre pays porte à l'échelle internationale sont une bonne chose, il faut aussi à l'échelle européenne, se battre pour que la loi sur le devoir de vigilance des grandes entreprises puissent trouver un débouché et notamment aller dans le sens de la mise en oeuvre une directive qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des pays européens, merci. Merci monsieur Marie. L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Annick à la ministre du Travail, la parole est à madame Annick millions. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues permettez-moi d'attirer votre attention, monsieur le Ministre sur la perte pour les territoires des services rendus par les structures médico-social et les associations relevant du secteur marchand, à la suite du gel des contrats aidés, certes, une réforme du dispositif devenait nécessaire mais depuis son annonce brutale, le manque de visibilité des mesures palliatives du gouvernement suscitent l'inquiétude en la matière, il est à craindre que les solutions attendues de la mission relative à l'innovation sociale au service de la lutte contre l'exclusion du marché du travail confié à Jean-Marc Borel au laisse de côté, nombres d'employé précaires, peu susceptibles de se former si les études à l'encontre du dispositif ne sont pas à mettre en doute, il conviendrait de ne pas occulter l'observation des économistes selon laquelle rien ne permet d'imaginer les conséquences de leur disparation disparition sur l'emploi avec le gel des contrats aidés, pas déjà touchée par la diminution des crédits accordés aux établissements publics accueillant les personnes âgées seront contraints de poursuivre la réduction de leurs effectifs alors que le bien être et la sécurité de nos aînés sont déjà très dégradée, les pas de pardon Tom hier de Longeville-sur-Mer s'est vu refuser le renouvellement d'une collaboratrice à un poste essentiel sans solution alternative, les nouvelles modalités de subventions ouvre également de sombres perspectives pour l'Union générale des Pays de Loire qui accompagne, plus de 53000 jeunes par an sur le territoire, précisément, 6 jeunes sur 10 sont considérés comme en sortie positive après 3 ans plus de 1300 contrats d'avenir ont été signés fin août 2017 entre jeunes et employeurs de même les restrictions déstabilise le fonctionnement des employeurs associatifs dont la réussite en matière d'insertion professionnelle n'est plus à démontrer, la Fédération de Vendée, de la Ligue de l'enseignement ne pourra plus gérer la continuité d'activités sociales et culturelles avec un déficit de dizaines d'emplois aidés autre effet pervers, les responsables de certaines de ses structures, se retournent vers les maires en désespoir de cause, pensant que celles-ci vont pouvoir les secourir, alors même que les Budgets des collectivités sont de plus en plus contraint le cas s'est posé pour les associations d'accueil et de protection des femmes en détresse en Vendée également alors que c'est la grande cause du quinquennat égalité hommes-femmes a été annoncée il y a peu le maillage associatif participe à l'équilibre social de notre territoire auquel le Sénat est fondamentalement attaché aussi notre commission de la culture, a-t-elle lancé une mission d'information visant l'impact de la réduction des contrats aidés sur le secteur associatif, me référant à la sacralisation des contrats aidés du secteur non marchand sur l'impulsion du président de la République, je vous serais gré de nous préciser, madame, monsieur, pardon le ministre si un moratoire d'un an seraient envisageable pour les structures médico-social et les associations relevant du secteur marchand, merci, c'est un peu long, merci. Si Madame Bignon tout à fait dans les temps, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, madame la présidente, madame la sénatrice, ça me rappelle quelques souvenirs avec la commission des affaires sociales, et cette loi travail dont j'avais été corapporteur que de porter la réponse de ma collègue, Muriel Pénicaud, qui malheureusement est retenue et et aurait souhaité pouvoir vous répondre plus directement, on est tous sur notre territoire bien attaché à l'action, effectivement, notamment des associations que vous évoquez, d'aide à domicile ou de soins à domicile sans lesquels je crois qu'un certain nombre de personnes auraient du mal à pouvoir hé bien rester, rester à domicile, or cette naturellement un axe prioritaire effectivement, le gouvernement a fait le le choix de d'orienter sa politique d'insertion durable à la vers les publics qui sont le plus éloignés de l'emploi et également pour les insérer dans le secteur marchand, donc c'est ainsi que prioritairement les les contrats aidés, programmée en 2018, pour un montant d'1,45 milliard d'euros, hé bien seront recentrés sur le le secteur non marchand non marchand d'autant plus important que voilà, avec la reprise des opportunités peuvent peuvent voir le jour, alors pour autant, les contrats aidés, voilà pour être mobilisés par des employeurs qui mèneront une une véritable politique d'accompagnement ciblé de formation car elle donne plus d'atouts de capacité aux bénéficiaires pour s'insérer durablement dans dans l'emploi, il y a le grand plan d'investissement qui prévoit un montant de 15 milliards d'euros sur ce volet formation et vous l'avez évoqué une mission est confiée à Jean-Marc brûle au président du groupe SOS une entreprise exemplaire en matière d'économie sociale et solidaire, il justement qui vise à apporter des solutions d'insertion innovante, et donc cette à l'occasion de la présentation des conclusions de cette mission que hé bien le pourront être exploré un certain nombre naturellement de de mesures pour l'avenir, mais d'ores et déjà, je veux rappeler que le secteur médico-social et les associations bénéficieront de l'action du gouvernement en faveur de la baisse du coût du travail, puisque le crédit d'impôts, de taxes sur les salaires, hé bien s'élèvera à 600 millions d'euros en 2018 et en 2019 à 1 milliard 4 de baisses de charges parce que, on le sait, parfois les équilibres financiers sont précaires dans ce type d'association et il faut tout faire pour que, en tous les cas, leurs activités et leur pérennité ne soit pas remise en cause, c'était en tous les cas un attachement que nous partageons avec vous c'est vrai. Merci monsieur le ministre de la parole est à madame Annick Billon pour répondre au ministre. Merci Madame Laberge présidente merci Monsieur le Ministre, ce que je déplore, essentiellement, c'est la méthode, en réalité, on nous annonce la suppression des contrats aidés au niveau des associations et je crois que, aujourd'hui, les associations se retourne, à juste titre, vers les collectivités qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens d'assumer les fonctions, on a mis en place d'étape une obligation faite par l'État au niveau de l'éducation, c'est font intervenir, nombre d'associations qui, de ce fait on pu embaucher des contrats aidés, on leur supprime donc je crois que certaines missions sont des missions qui doivent être assurés non pas par les associations, mais par le service public, donc Monsieur Blanc les ministres flanker et Madame Cluzel ont annoncé, hier, concernant les assistants de vie scolaire, plus de formation plus d'accompagnants, beaucoup d'annonces, moi je souhaite voir ces annonces traduite dans les faits maintenant sur le terrain puisque les associations et les notamment les associations qui protège les femmes sont dans l'attente de ces mesures parce que, on le voit pour la protection des des femmes qui, qui subissent des violences, c'est bien souvent les associations qui font le travail, merci. Merci madame Guillon. L'ordre du jour appelle à questions orales de Monsieur Guillaume Gontard au Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, la parole est à monsieur Guillaume Gontard. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, vous annonciez le 20 septembre dernier à la fin des aides au maintien de l'agriculture biologique, précisant qu'il revenait désormais au marché de soutenir le maintien à ce type d'agriculture, nous aurions pu croire à une annonce du porte-parole de la FNSEA, je vous l'avoue, c'est un très mauvais signal envoyé un secteur dynamique de notre économie, les bienfaits pour l'environnement ne sont pas à démontrer cette annonce est contradictoire avec votre volonté de parvenir à 8 pourcent de surface agricole utilisable exploitée en bio à l'horizon 2020, vous me répondrez que cet argent est intégralement transférée aux aides à la conversion mais ces aides ne couvre qu'une période de 5 ans, alors qu'il faut en moyenne 6 à 7 ans pour qu'une nouvelle exploitation bio se stabilise et devienne rentable, c'était tout l'objet des aides au maintien que vous supprimez ceci est d'autant plus incompréhensible que les aides au maintien de la créature conventionnels sont conservés concentre 85 96 pourcent des aides à l'agriculture, de surcroît, ce financement de l'État permettait de débloquer l'aide européenne fait avec un mécanisme particulièrement avantageux puisque chaque Euro dépensé par Paris correspondait à 3 euros dépensés par Bruxelles ainsi ce sont 6 à 8 millions d'euros d'aide au maintien que ne feront pas les jeunes exploitations biologiques et potentiellement 4 fois plus en effet avec ce désengagement de l'État vous confier aux seules régions et aux abords des agences de l'eau déjà exangue la responsabilité d'apporter l'intégralité de la contribution publique nationale au fait même dans les régions en pointe sur le bio, cet effort financier semble impossible : dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes c'est une catastrophe qui s'annonce, la région de contribuer pas au fait adhère ne compensera certainement pas l'Delagrange, de l'État, ainsi, c'est une perte sèche de plusieurs millions d'euros pour la 2ème, région qui compte le plus d'exploitations bio dans le pays. Monsieur le ministre, le président de la République a annoncé, dans le cas des états généraux de l'alimentation, la mise en place d'une enveloppe de 200 millions pour financer la transition agricole, pouvez-vous nous dire quels en sont les objectifs actuels interprofession seront-elles confiées avec quel pluralisme syndical et enfin créer proportion sera-t-elle ou directement à l'agriculture biologique, je remercie. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, je vous laisse d'abord la responsabilité de l'entame de votre de votre question et je vais vous réponde précisément et essentiellement sur le sur Comme il se doit, les aides à l'agriculture biologique, vous le savez, sont des dispositifs du second pilier de la PAC, qui permettent d'accompagner les agriculteurs dans la transition vers des systèmes agricoles conciliant à la fois performance économique, social, environnemental, l'État mobilise des moyens particulièrement importants pour le financement de ces dispositifs et le budget total sur 2014, 2020 pour les aides au bio a été multiplié par 3 par rapport à la programmation 2007, 2013, ses soutiens à l'agriculture bio ont été particulièrement efficaces et ont permis un fort développement, vous savez de ce mode de production ces dernières années avec 1,5 millions d'hectares en bio 30 2000 exploitations et 15000, transformateurs et distributeurs qui ont été recensés en 2016 le soutien même doit maintenant porter en priorité sur la conversion à l'agriculture biologique, afin que la production française soit en rendez-vous avec la forte demande des consommateurs, l'enjeu est aussi de relever le défi de proposer 50 pourcent d'alimentation biologique ou sous signe officiel de qualité dans la restauration collective, conformément aux engagements du président de la République pour autant l'aide au maintien n'est pas supprimée, on ne sait pas dans quelle langue va pouvoir le dire un jour, mais l'aide au maintien n'est pas supprimer ce dispositif

ici davantage de crédits mobilisés et consacré à l'agriculture biologique, l'État continuera bien évidemment à financer les engagements en maintien qui ont été souscrits avant 2018 jusqu'à leur terme, ces aides étant attribuée pour une durée de 5 ans, et vous le savez, les autres financeurs, en particulier les collectivités, les agences de l'eau pourront continuer à financer de nouveaux engagements en matière de maintien et en complément de ces aides, un crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique et prorogé et revalorisée afin d'assurer un soutien Simple pérenne et uniforme à l'ensemble du territoire, le fonds d'avenir bio est par ailleurs maintenue, qui permet aussi de soutenir des projets de structuration de la filière bio avec un important effet de levier, vous voyez, Monsieur le Sénateur, l'État reste attentif sur cette question sur la dynamique de développement du bio, de l'agriculture pour les prochains mois et et pour les prochaines années, merci. Si Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Guillaume Gontard pour répondre à Monsieur le Ministre. Merci monsieur le ministre, moi si je suis, je suis d'accord sur le constat que vous faites au début de votre intervention, permettez-moi d'avoir un petit peu des doutes sur sur votre sur votre développement puisque bah, vous confirmez que les aides sont sont bien sur 5 ans et que sur ce type d'agriculture, on a besoin de d'avoir un soutien beaucoup plus : ensuite vous vous flécher les aides sur les sur les régions, mais je pense qu'on risque d'avoir une vraie distorsion entre les régions entre des régions qui ne souhaiteront pas ou qui ne pourront pas abonder et se substituer à l'État sur le sur le fond et sur le le fond sur cette cette agriculteur bio, on est aujourd'hui sur la journée mondiale des sols et je pense qu'il faut revoir notre notre fonctionnement de de penser notre manière de penser et notre lien avec avec

pour les agriculteurs, je dirais, surtout pour les agriculteurs parce que, au bout de la chaîne, c'est eux qui subissent directement ce je dirais ce ce ce mauvais cercle à la fois financièrement puisque il s'endette mais aussi en matière de santé parce que tous ces produits, c'est quand même qui qui en subissent les conséquences directes, je pense qu'il est réellement tant d'agir, j'ai entendu ce que vous m'avez dit mais je vous encourage vivement à aller encore plus loin, parce qu'il me semble que c'est la une, la seule solution, merci Monsieur. Si chers Si chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de madame Pascale Borie au Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, la parole est à madame pourri. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, la sécheresse que subissent de nombreux départements français et tout particulièrement le garer sans précédent, nous ne sommes qu'au début d'un phénomène qui aura indéniablement des répercussions sociales fortes avec mes collègues au Sénat et Assemblée nationale, nous avons déjà pu vous présenter les dégâts en cours à ce sujet sans avoir, hélas, pour l'instant de réponse satisfaisante, en effet, avec 25 jours d'avance, la récolte a été la plus faible depuis 1945 la baisse de rendement atteint de 25 à 30 pourcent dans le département, avec des pics à plus de 40 pourcent pour les du Rhône gardoise, le secteur dont je suis élue locale mais la sécheresse n'entraîne d'autres effets dont l'ampleur n'est pas encore totalement saisissable, on assiste à une mortalité sans précédent des 7 plus particulièrement des Plantier et dans certains secteurs proches de la mer à des remontées de sel inquiétante aussi, les agriculteurs vont subir une baisse tendancielle sur plusieurs annuité de la production de vin non compensée par la hausse des prix, vins de pays comme les vignobles classés en AOC, à l'instar des du Rhône du Tavel, ou encore des Costières de Nîmes vont souffrir de cette crise, la souffrance est grande chez ces agriculteurs, à cela s'ajoute l'importation illégale des vins étrangers et la concurrence déloyale de certains pays européens qui ne respectent en rien les mêmes et que nos viticulteurs une distorsion devenue encore plus criante avec la décision de votre goût et gouvernement d'anticiper l'interdiction du glyphosate, nous ne pouvons rester sans rien faire, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux doit pouvoir aider cette agriculture qui est au coeur de l'identité de la France au-delà du fond spécifique de 30 millions d'euros, ou la mise en place d'arrêtés de catastrophe naturelle anus, nous demandons des décisions fortes pour pouvoir mieux travailler, comme par exemple un soutien au cas des coopératives à partir d'un seuil de perte ainsi une prise en charge des pertes de fond sur Plantier un étiquetage clair et lisible la provenance sur le vin en vrac, trop souvent, la France va plus loin que ce qui est recommandé par les directives, ce qui alourdit les coûts de production de prône aux agriculteurs le débat lyrique de l'irrigation doit être enfin poser mon département des bénéficie de l'eau du canal du Rhône néanmoins tout le Gard n'a pas accès à cette irrigation et la question se pose pour d'autres départements nous devons élargir les possibilités d'irrigation et crée un schéma régional, voire national pour accroître le potentiel en eau grâce notamment à la création de retenues ou l'utilisation des eaux usées, traitées comme cela est autorisé dans d'autres pays européens, les étés seront de plus en plus chaud, monsieur le Ministre, je vous demande donc de prévoir de nouvelles mesures pour ses agriculteurs et d'entamer une réflexion sur le long terme pour prévenir ces phénomènes de sécheresse, je vous remercie. Merci Madame la parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, je connais bien la situation que vous vivez dans le dans le Gard après tous ces mois sans sans eau de pluie pour venir irriguer vignes, j'ai rencontré une délégation de viticulteurs gardois, la semaine dernière lors du du site qui ont eu l'occasion de me de me rappeler la détresse qui était la leur et que j'ai parfaitement entendu et c'est vrai qu'au cours de l'année 2017 la filière viticole a été sévèrement touchée par des nombreux phénomènes et dans notre département, les estimations nationales anticipe une récolte de de 20 pour 2017 de 36,8 millions d'hectolitres, soit 19 pourcent de moins que 2016 et le volume prévisionnel de la récolte 2017 c'est lève 2 67 millions d'hectolitres, soit une baisse significative de 20 2 7 pourcent par rapport à la campagne précédente, dans ce contexte de dahlias multiples des mesures conjoncturelles ont d'ores et déjà été déployés, madame la sénatrice par les services de l'État pour accompagner les exploitations viticoles, qui ont été sévèrement touchés autour de au cours de cette campagne de 2 phénomènes climatiques le dégrèvement, pardon, de la taxe sur le foncier non bâti, la prise en charge des cotisations sociales pour un montant de 30 millions d'euros, la mise en place de mesures d'allégement des charges financières ouverte jusqu'au 31 décembre 2017 et accessible aux viticulteurs, par ailleurs, j'ai souhaité dernièrement la mise en place de cellules pour identifier les problèmes spécifiques et ces cellules identifieront étudieront de manière confidentielle, les différentes situations pour orienter les exploitants vers les dispositifs qui seront les mieux adaptés pour chacun d'eux mêmes et face à la multiplication des crises qui touchent le secteur agricole et le secteur viticole mes services ont engagé des travaux pour développer une approche globale de la gestion des risques et cette approche globale, madame la sénatrice, elle devra viser à adapter les outils à la gestion des aléas et notamment s'intéresser à des propositions formulées pour la la mise en place de d'une épargne de précaution ou l'amélioration de la dotation pour aléas et puis, l'agriculture est un des secteurs particulièrement exposés aux modifications hydrologiques et nous avons précisé lors d'une d'une communication le 9 août dernier des orientations précises en matière de gestion durable de l'eau autour de 2 objectifs, encourager la sobriété des usages et réguler en amont la ressource pour faire émerger dans l'ensemble du territoire des solutions adaptées adaptées aux besoins et aux contextes locaux, cela passe par la réalisation là où c'est utile, la hausse est durable, 2 projets de stockage hivernale de l'eau pour réduire les prélèvements en période sèche et éviter l'augmentation des prélèvements estivaux dans les zones qui sont menacés par les changements climatiques, ces orientations feront l'objet de déclinaison opérationnelle dans les mois à venir, et j'en termine, vous constaterez avec moi madame la sénatrice que ces aides ponctuelles, les allégements de charges, l'épargne de précaution, la dotation pour aléas et la gestion de l'eau, c'est une stratégie complète au service de la viticulture et au service de votre département, je vous remercie. La parole de Madame Pascale Borie pour répondre à Monsieur le Ministre. Oui monsieur, ministre, je vous remercie, je vous écoutez je vous remercie d'avoir pris le temps de justement d'étudier cette situation délicate à laquelle se retrouvent confrontés les viticulteurs et de mettre en place cette cellule de réflexion à laquelle je ne doute pas, vous, ce vous serez associé les viticulteurs, je crois qu'il est important effectivement d'avoir une vision à long terme, je vous ai fait part donc de certaines propositions et notamment sur ce schéma de de réflexion de schéma régional, voire national d'irrigation et avec des possibilités d'utilisation aussi des eaux usées traitées, je crois que ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre que la souffrance d'aviculture des viticulteurs soit trop criantes car vous le savez très bien, en fait, la crise viticole, ça en fait s'accompagne de conflits violents et nous ne pouvons pas aller jusque-là. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Dominique Vatrin transmise à la garde des Sceaux, ministre de la justice, la parole est à monsieur Maître. Madame la présidente, monsieur le Ministre, vous le savez, dès son installation à la tête du gouvernement, j'ai écrit au 1er ministre au sujet du dossier des mineurs grévistes 48 et 52 injustement licencies aujourd'hui bien du chemin reste encore à parcourir par l'État pour une réhabilitation complète, en effet, bien que la République est reconnu officiellement leur préjudice depuis plusieurs années maintenant, à ce jour, seuls 36 dossiers de mineurs ont pu bénéficier des nouvelles dispositions dispositions des lois de finances pour 2015 et 2017, tandis que 41 d'entre eux devaient pouvoir-ils être éligible, il reste 150 cas identifiés, qui surfe, 70 ans après les événements, caractère fermé de la loi de finances pour 2005, les enfants d'droit 4 décès de leurs parents ne peuvent en effet avoir recours aux indemnisations prévues par la loi de prix finance pour 2005, ni donc aux indemnisations proposées en 2015, une fin de non-recevoir que les intéressés vivent légitimement comme une discrimination une ségrégation sur la question du droit, l'ancien garde des sceaux Madame Taubira fait son possible, mais sans mise en oeuvre des moyens nécessaires sur l'implication des autres ministères concernés du fait du mépris affiché par l'ancien garde des Sceaux Monsieur Urvoas s', la situation n'a plus évolué, le dossier semble même aujourd'hui au point mort, si j'en juge par la non réponse du 1er ministre à mon courrier du 29 mai 2017 dans lequel j'évoquais le long combat mené par ses victimes et le syndicat CGT mines à l'instar d'ailleurs de Norbert Gilmez, fer de lance de cette lutte, aujourd'hui âgée de 96 ans, décoré de la Légion d'honneur mais qui attend lui aussi une réparation complète, monsieur le Ministre, le temps presse, les mineurs pour la plupart d'anciens résistants à l'occupation nazie, se sont battus pour leurs droits sociaux et ont été lourdement condamnés, assimilés à des terroristes, ils ont été réprimées puis licencié chasser avec la fin de leur famille, de leur logement, des écoles des mines de leur ville lors épouses et leurs enfants ont beaucoup souffert après les attentes et les espoirs déçus : quelles mesures comptez-vous inscrire dans le PLF 2018 ou dans un proche et le prochain budget rectificatif pour rendre justice aux mineurs et à leurs familles, comment comptez-vous permettre aux filles et fils de mineur, eux-mêmes victimes d'accéder aussi au dispositif en cours : avez-vous la volonté de réparer ce terrorisme d'État, par exemple en faisant bénéficier ces mineurs d'une reconstitution de carrière en application de la loi d'amnistie de 1980 comme cela était le cas des fonctionnaires concernés. Merci monsieur Vautrain, la parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, voudrait bien excuser ce matin, l'absence de ma collègue Garde des Sceaux ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui est en grande déplacements actuellement à Nouméa avec le 1er le 1er ministre vous avez appelé l'attention du. Même sur la question de l'indemnisation des mineurs grévistes de 1948 et 1952 amnistiés par la loi du 4 août 1980 où l'avait rappelé à l'initiative personnelle de Christiane Taubira, le gouvernement a été à l'origine d'un amendement, devenu l'article 100 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 par lequel la République reconnaît solennellement : d'une part le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour fait de grève des mineurs grévistes en 1948 et 52 et d'autre part, les atteintes portées à leurs droits fondamentaux et les préjudice en résultant, à ce titre, la loi a ouvert aux mineurs dont les dossiers avaient été antérieurement instruit par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en application de l'article 107 de la loi de finances pour 2005, du 30 décembre 2004, le bénéfice d'une allocation forfaitaire d'un montant de 30000 euros pour chacun des mineurs concernés ou leur conjoint survivant une allocation complémentaire spécifique de 5000 euros, a été également prévues au bénéfice Direct de chaque enfant de séminaires, les demandes de bénéfice des allocations devrait être adressées avant le 31 décembre 2015 Allen j'ai DM chargé de garantir au nom de l'État, l'application des droits sociaux et des prestations des anciens mineurs, l'agence a instruit l'ensemble des dossiers qui lui ont été adressées avant cette date, au vu des informations qui lui ont été communiquées, elle a versé à cette mineurs et 15 conjoint survivant, ainsi qu'à 97 enfant les allocations prévues par ce dispositif, pour un montant total de 1 virgule 6 46 millions d'euros, soucieux de voir examiner les dossiers qui n'aurait pas été adressées avant le 31 décembre 2015, le gouvernement a souhaité proroger jusqu'au 1er juin 2017, la date limite de dépôt des demandes de bénéfice du dispositif d'à l'occasion un amendement en ce sens, a ainsi été votée dans le cadre de la loi de finances rectificative, la loi de finances de 2015 a également prévu que les mineurs bénéficiaires des prestations chauffage et de logement en espèces prévues par le statut minier ou le conjoint survivant peut faire valoir auprès de l'agence tout élément qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ses prestations, il appartient ici aux intéressés de faire valoir ces éléments auprès de l'agence, qui relève de la double tutelle du ministère de l'environnement et de l'énergie et du ministère de l'Économie et des Finances, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, la parole est à monsieur Dominique va Vautrin pour répondre à Monsieur minute. qu'aucun ministre de tutelle, concernés par ce dossier ne soit présent sur le banc du gouvernement, pour répondre aux filles et fils de mineur à qui est toujours refusé le bénéfice de l'indemnisation au prétexte que leurs parents sont décédés, or sur ce point vous n'avait apporté aucune avancée, ni aucune réponse même 2ème non répond sur l'application de la loi d'amnistie de 81 je vous rappelle quand même sur ce point que les généraux félons de l'OS ont obtenu une reconstitution de carrière une indemnisation complète, c'est quand même un comble que des mineurs qui ont pour beaucoup participé à la libération de notre pays du joug fasciste et qui n'ont pas épargné le receveur au sortir de la sortir de la guerre contre les nazis et qui ont donc permis de redresser notre pays en soient exclus d'ailleurs, il y avait dans la loi d'amnistie une clause d'indignité qui ne peut valoir de refus maintenant puisque ces mineurs ont été officiellement réhabilité par la République, alors moi je poserais pour terminer une question : c'est qui s'occupe du dossier, vous avez évoqué plusieurs ministères effectivement les ministères de tutelle, l'environnement, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de la justice, moi je pense que il serait judicieux que ce soit le 1er ministre lui-même qui se saisissent de ce dossier afin que on se renvoie pas la balle et qui a une véritable volonté politique affichée il y a besoin d'un signal politique fort au plus haut niveau de l'État pour règlement pour le règlement définitif de ce contentieux, c'est le message que je voulais vous faire passer Monsieur le Ministre.

de Madame la Ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, puisque ma question concerne l'engagement présidentiel de construire 15000 places de prison en 5 ans ma question est très précise : premièrement, je souhaite savoir si vous pouvez me confirmer que cette programmation intègre bien le plan de 3200 places annoncées par Madame Taubira pour la période 2015, 2017, mais aussi celui annoncé en février de cette année, portant une première liste de 33 établissements, pour un total de 3900 places supplémentaires si je demande ces précisions c'est parce que le nouvel établissement de Lure sonne était inscrit dans le programme Taubira 2015, 2017, à la suite de la fermeture de la maison d'arrêt dure le 14 septembre 2015, a eu un grand moment Olson, on a eu un comité interministériel délocalisé, avec la présence du président Hollande que vous avez servi à cette époque et qui a d'ailleurs confirmé cet engagement de l'État lors de ce comité interministériel, donc c'est important cette parole, je souhaite savoir si les crédits nécessaires à la réalisation des travaux tant en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement bien sûr seront bien inscrits dans la première programmation du plan de 15000 places et je souhaite également être éclairés sur la réalité de la fonctionnalité de cette, de ce nouvel établissement qui était prévue, à une époque de 300 places maintenant 250 donc est-ce que ce sont uniquement des nouvelles places un assemblage de nouvelles places de remplacement d'autres établissements, à commencer par celui de Vesoul 2ème maison d'arrêt de Haute-Saône, que nous ne souhaitons pas voir disparaître pour une raison simple, pas pour des raisons archaïque de maintenir tout ce qui existe, mais tout simplement parce que l'État, au pied du tribunal et qu'on sait très bien quand on ferme une maison d'arrêt, on risque de fermer le tribunal, peu de temps après, donc on souhaite absolument garder cette maison d'arrêt de Vesoul, merci Monsieur le Ministre, de bien vouloir m'éclairer. Merci monsieur raison : la parole est à monsieur ministre de l'Agriculture et de l'alimentation Monsieur. Stéphane Travert. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Michel Raison, je vais essayer à travers 13 la réponse à cette question, d'être le plus précis possible sur la demande que vous que vous formulez et je vous prie, une nouvelle fois d'excuser ma collègue collègue Nicole Belloubet Garde des Sceaux ministre de la justice pour son absence étant retenu avec le 1er ministre en Nouvelle Calédonie et donc vous avez souhaité appeler l'attention de Madame la Garde des Sceaux sur cette question de la construction de la maison d'arrêt de de Lure, le président de la République avait pris l'engagement de créer 15000 places de prison supplémentaires pour atteindre l'objectif de l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt où la très forte peuvent surpopulation carcérale aujourd'hui dégradent la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires, le programme 15000 prévoit notamment la construction sur la période 2018, 2027, une trentaine de maisons d'arrêt et de centres pénitentiaires, ainsi que d'une quinzaine de quartiers de préparation à la sortie, certaines de ces opérations, qui relevaient de programmes antérieurs comme le programme 3200 auquel vous avez fait référence seront intégrés à cette programmation l'ensemble des opérations qui avaient été identifiés ces derniers mois, font actuellement l'objet d'études de faisabilité, partout où où des terrains ont été proposés ou de recherche foncière, là où les investigations n'ont pas permis encore d'aboutir et c'est au vu des résultats de l'ensemble de ces travaux que la liste des opérations retenues sera arrêté dans les tout prochains mois, elle sera annoncée dans le cadre de la loi de programmation pour la justice que la garde des Sceaux présentera au Parlement à la fin du printemps 2018, à ce stade, aujourd'hui encore trop tôt pour se prononcer sur telle ou telle opération dans la mesure où les expertises techniques et les consultations en particulier avec les élus locaux se poursuivent, le choix des implantations sera de toute façon, guidée par les besoins pénitentiaire les ressources budgétaires et les conditions d'accueil des futurs établissements je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, j'accepte évidemment d'excuser Madame la Garde des Sceaux, faut bien qu'elle fasse son travail, à l'extérieur de la métropole, mais la réponse n'est pas très précises parce que les travaux préparatifs et la mise à disposition de terrains par les collectivités fait donc j'aurais souhaité qu'on puisse me dire si à partir de moment où cette période était passé, on pouvait effectivement compter sur la construction de ce nouvel établissement, vous m'avez dit du moins, on vous a fait dire que certaines relèvent du plan 3200 mais je sais toujours pas si eurent fait partie des certaines elle est dedans, donc c'est déjà quand même une première précision, mais j'aurais souhaité qu'on puisse me dire oui, puisque les études techniques sont terminées les études environnementales sont terminés, le terrain mis à disposition par la la commune de l'UE, donc on au Jaurès souhaité qu'on puisse me dire aujourd'hui fermement oui ce dossier bien retenu, donc j'ai encore une incertitude, donc on reviendra dans peu de temps, poser la question, merci. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Yannick Vaugrenard à la ministre des solidarités, de la santé, la parole est à monsieur Yannick Vaugrenard. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en octobre 2012 François Hollande annonçait la généralisation à horizon 2017 de l'accès à une couverture complémentaire santé de qualité, en juin 2015 au congrès de la Mutualité, à Nantes, le président de la République avait indiqué ne pas avoir oublié les personnes retraitées avec une généralisation de la complémentaire santé effective d'ici 2017 cependant, cela n'a pas été fait, la situation a même empiré puisque les retraités sont victimes aujourd'hui d'une triple peine : baisse du revenu perd cofinancement de leurs cotisations par leur employeur et pertes des aides fiscales, en moyenne, ils voient leur complémentaire santé multipliée par 3 et demi, passant de 283 à 998 euros par an sur la problématique particulière des soins optiques une étude estime que les retraités cumule les inconvénients, ils ont les besoins les plus élevés en terme d'optique médicale et paient l'intégralité de leurs cotisations, une paire de lunettes leur revient à 400 euros tandis que la plupart des actifs sont remboursés par l'assurance maladie et leur complémentaire santé auteur souvent de 100 pourcent le gouvernement précédent s'était engagé à encadrer fortement les hausses de cotisations aux complémentaires santé pour les retraités, cependant, le décret paru en mars de cette année, limite l'augmentation possible des cotisations sur 3 ans, laissant une liberté totale aux mutuelles, à partir de la 4ème année de retraite, il était également courant que les retraités soient pénalisés par des augmentations brutales des tarifs de leur mutuelle, passé un certain âge, elles attirent ceux de 60 ans, avec un tarif à 50 euros mais il pas soudainement à 100 euros lorsqu'ils atteignent 70 ans, l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, porte précisément sur les frais d'optique dentaire et de prothèses auditives avec l'engagement d'arrêt, ça charge nulle sans augmentation du prix des mutuelles cette promesse sera-t-elle tenue le sera-t-elle pour tous, y compris pour les retraités, madame la ministre, pouvez-vous nous détailler les mesures que compte prendre le gouvernement pour soutenir les retraités dans leurs dépenses de santé, un système de crédit d'impôt couvrant la hausse des cotisations nouvelles à partir de 70 ans pourrait-il par exemple être mise en place, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre de la solidarité, de la santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Vaugrenard merci pour vous, lunettes, madame la sénatrice, qui me permet de répondre à la question du sénateur, le gouvernement a parfaitement conscience évidemment des difficultés que peuvent rencontrer les retraités pour accéder à une complémentaire santé abordable, l'aide à la complémentaire santé permet de tenir compte de l'augmentation des primes avec l'âge, cette aide est nettement plus élevé pour les personnes âgées de plus de 60 ans, son montant s'élève à 550 euros contre 350 euros pour les personnes de 50 à 59 ans, pour les anciens, salarié du secteur privé, le décret du 21 mars 2017 renforce les garanties et a ainsi permis de lisser les 3 premières années postérieures à la fin de l'emploi dans l'entreprise, ainsi que l'augmentation tarifaire par les assurés, au moment de leur départ à la retraite pour les retraités de la fonction publique, le dispositif de référencement de conventionnement de labellisation tiennent compte de critères de solidarité envers les plus âgés, et notamment des transferts entre générations, ce qui permet d'assurer une véritable mutualisation au-delà de ces dispositions le gouvernement porte une attention particulière aux personnes âgées, les plus modestes, il est prévu dans le PLFSS 2018 une revalorisation exceptionnelle de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui s'élèvera à 903 euros, soit 100 euros supplémentaires dès janvier 2020 pour une personne seule, pour préserver l'accès à une complémentaire santé aux plus modestes, j'ai souhaité prévoir un abattement sur les montants de l'Aspa et de l'allocation adulte handicapé, pris en compte pour évaluer les revenus pour l'accès à la couverture universelle maladie complémentaire de la CMU-C et à l'aide au paiement d'une complémentaire santé, cette disposition permettra ainsi à plus de 50000 personnes à revenus très modestes, de continuer à bénéficier de la CMU-C et de laisser enfin vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, le gouvernement travaille actuellement à la mise en place d'un reste à charge nulle sur l'optique l'audio-prothèses et des soins dentaires bien évidemment couvrant les personnes âgées, quelle que soit leur âge, afin de permettre l'accès de tous à des soins de qualité et ces évolutions permettront notamment pour les personnes âgées, un meilleur accès aux soins sans reste à charge, je vous remercie. Merci madame la ministre, la parole est à monsieur Vaugrenard pour répondre à Madame la Ministre. Oui, merci, Madame la Ministre, de bien voir de bien avoir voulu répondre à nos interrogations et mes propositions, je suis perplexe, vous nous dites à la fin de leurs interventions, le gouvernement met à l'étude la possibilité de rembourser totalement les soins d'optique, les soins dentaires, en particulier, voire avoir auditif, mais c'est, c'est à l'étude, donc j'espère que les choses vont vont avancer le le plus rapidement possible, par ailleurs, vous faites état dans votre réponse, des propositions qui qui sont faites, notamment dans le PLFSS de soutien supplémentaire aux personnes âgées en difficulté importante je vous donne acte bien sûr de cet effort qui est fait et je pense que c'est un élément incontestablement positif par rapport aux mutuelles complémentaires santé au début de son intervention, vous nous avez dit que l'augmentation était ne pouvait pas être possible durant les 3 premières années qui suivent 60 ans qui suivent la retraite sauf que très souvent et je le dis dans ma précédente intervention les mutuelles à 60 ans donne un tarif de 50 euros à 70 ans, il double la mise, Santoro ce qui pose un problème extrêmement important en terme de de coûts à supporter par les personnes qui n'est pas ce qui n'est pas ce que 70 ans la santé a un coût, considérons globalement, quelle qu'elle n'a pas de prix que la solidarité intergénérationnelle doit être doit être importante, d'autant plus que de plus en plus dans les familles, les personnes retraitées aident aussi les jeunes en difficulté, c'est un élément qui n'existaient pas ou peu voici 20 20 ou 30 ans, enfin Madame Denis je voudrais refaire la proposition que je vous ai fait tout à l'heure, un système de crédit d'impôt qui pourrait permettre de couvrir Les hausses de cotisations des complémentaires santé à partir de 70 ans, je souhaite que ce 1er véritablement ce soit une piste qui se regarder avec attention par le gouvernement et par vous-même, Jean d'Ormesson, nous a quitté cette nuit pas de même bord politique, moi je retiens une de ces phrases, ce qui est clair, dit existence et d'espérance, j'espère, Madame la Ministre, que vous prendra en compte les propositions que je vous ai fait. Si chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Catherine Procaccia, au ministre de l'Économie et des Finances, la parole est à madame procréation. Merci madame la présidente, madame la secrétaire d'État mais, chers collègues, j'ai souhaité par cette question, attiré l'attention de monsieur le ministre de l'Économie et des Finances sur les vols et les attaques aux distributeurs automatiques de billets, ces attaques lors d'un retrait à un distributeur de billets donnant sur une rue se multiplient selon un mode opératoire bien connu des services de police et des banques, ces vols sont observés sur l'ensemble du territoire et très très régulièrement à Paris, la procédure est la suivante, et j'en profite pour attirer l'attention de tous sur cette procédure après avoir inséré la carte bancaire, le titulaire tape son code personnel mais avant d'avoir eu le temps de choisir le montant de son retrait, surgit un ou plusieurs individus alors que le réflexe malheureusement et de tenter de protéger la carte de crédit, les voleurs bouscule avec plus ou moins de violence, la personne se place devant le distributeur de billets et tape une somme souvent importantes sur le clavier, avant de prendre la fuite avec les espèces étrangement la carte de crédit n'est généralement pas dérobé, hélas pour le client qui n'est pas assurée et se retrouve avec un débit important sur son compte, parfois même avec un découpe et avec des agios, ma question est simple j'aimerais savoir comment vous entendez faire évoluer la protection des clients qui même prudent sont démunis face à la recrudescence de ce type d'attaque, les assurances incluses dans les cartes bancaires ne couvre pas ce type d'agression alors ma question est donc : le gouvernement prévoit-il de faire évoluer la réglementation à partir du moment où le vol éprouvés par des caméras de surveillance

madame la sénatrice Catherine Procaccia je vous remercie d'attirer notre attention sur ce type de vols et d'agressions ces situations mérite en effet d'être examiné dans le cadre de telles pratiques, le code a déjà été renseigné par l'usager, le client de la banque, cette situation et de ce fait problématique car elle ne semblent pas pouvoir bénéficier du régime protecteur prévue par le Code monétaire et financier suivant lequel le titulaire de la carte ne supporte une franchise limitée en cas de perte ou de vol, cette situation sera porté à l'attention de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations, des émetteurs de moyens de paiement des opérateurs de systèmes de paiement des associations de commerçants des assure d'entreprises et des associations de consommateurs, cet observatoire a la capacité de proposer des moyens de lutter contre les atteintes à la sécurité des moyens de paiement dans ce cadre, je serai attentive aux solutions que les acteurs pourront apporter à ce problème et en tirerait le cas échéant les conclusions pour que si, pour ce qui concerne la réglementation. Merci, la parole est à Madame Procaccia pour répondre à Madame la secrétaire d'État. Merci madame la présidente, madame, merci madame la secrétaire d'État, donc si je comprends bien, on va attendre la réaction de l'Observatoire de la sécurité et le gouvernement, éventuellement on pourra prendre un certain nombre de décisions ou pousser parce que c'est quand même assez illogique que ce soit le seul cas dans lequel le client n'est pas couvert la Audio 18 janvier je crois lorsqu'il y a vol de la carte bancaire à ce moment-là la franchise qui était de 150 euros va passer à 50 euros quand il y a des vols sur internet, on est remboursé par le biais d'Internet intégralement et le seul cas c'est quand on est attaqué aux distributeurs où on n'est pas couvert et même pas avec une franchise, donc j'espère effectivement que cette situation anormale sera prise en compte et je surveillerait de près ce que va dire l'observatoire et je je vous recontacterai où je saisirai le ministre de l'économie, c'est rien n'était fait, merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle à question orales de Madame Sophie taillé pour Lyon à la ministre du Travail, la parole est à madame taillé pour Madame la présidente, madame la ministre je souhaite interroger le gouvernement sur les conséquences pour l'exercice de la liberté syndicale, de la fermeture de plusieurs bourses du travail Evreux Villejuif Montigny Aubagne Tarbes Bobigny Châteauroux Béziers Nancy dans ces communes et dans d'autres la liberté syndicale est aujourd'hui altérée par des tentatives ou par l'expulsion des hébergements syndicaux des bourses du travail la liberté syndicale, bien que libertés fondamentales, protégées par le conseil constitutionnel en vertu notamment de l'annihiler 6 du préambule de la Constitution de 46 est régulièrement remise en cause dans les entreprises, on assiste à des sanctions, des mises à pied conservatoires des tentatives de licenciements de salariés protégés, bref la comment dirais-je, la, la, le dialogue social n'est pas toujours simple et les syndicats dénoncent un certain nombre de provocation et à ce mal être syndicale s'ajoute la remise en cause des hébergements syndicaux dans de nombreuses localités, c'est le cas à Villejuif où les organisations syndicales ont été sommés par la mairie de quitter la Bourse du travail, une telle décision prive les organisations syndicales de moyens d'exercer leur mission et prive aussi les salariés, notamment des petites, les toutes petites entreprises d'avoir accès à la formation syndicale pour défendent leurs droits lorsqu'ils sont isolés dans leur entreprise, le gouvernement annonce vouloir faire du dialogue et de la démocratie sociale une priorité de l'action du ministère du Travail, malheureusement la possibilité ouverte par les ordonnances adoptées récemment et qui doivent passer en 2ème lecture à la négociation directe dans les entreprises entre l'employeur et les salariés ne concourent pas vraiment alors l'organisation du travail ne peut se construire et s'appliquer sans la partition active la participation active des partenaires sociaux qui doivent jouer un rôle croissant dans sa conception et sa mise en oeuvre et pour ce faire, ils doivent avoir des outils compris des outils locaux au coeur des territoires et donc je vous demande si l'État entend garantir le maintien de ces bourses du travail qui sont souvent inscrite historiquement dans les territoires, y compris peut-être en participant financièrement garantissant juridiquement aux côtés des collectivités territoriales, à leurs frais de fonctionnement, surtout lorsque celle-ci rayonnent sur plusieurs communes alors qu'elle n'a pas que le budget que d'une seule, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Delphine Gény-Stéphann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Sophie par les polluants vous attirer l'attention de la ministre du Travail, sur les conséquences pour l'exercice de la liberté syndicale, de la fermeture de plusieurs bourses du travail un rapport de l'IGAS, remis en avril 2013 et suivie d'une autre en juillet 2015, a permis de constater que les mises à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales s'inscrivait dans un cadre juridique fragile et peu claire, fondée sur la notion d'usage, à quoi s'ajoutait des questions parfois complexe d'attribution des locaux et de répartition des charges d'entretien. C'est pourquoi un cadre juridique clair a été instaurée en 2016, ainsi les articles L 1311 18 et L 2144 3 du code général des collectivités territoriales, prévoit que les collectivités terreau écrite Royal ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à disposition des organisations syndicales, lorsque ces derniers en font la demande, cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention entre la collectivité et l'organisation syndicale. Par ailleurs, il revient désormais au maire, au président du conseil départemental au président du conseil régional au président d'un établissement public au local ou regroupant les collectivités territoriales ou au président d'un syndicat mixte de déterminer les conditions dans lesquelles l'usage de ses locaux peut-être proposé aux organisations syndicales à cet égard, le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d'administration de l'établissement ou ou du syndicat mixte déterminant tant que de besoin, la contribution du à raison de cette utilisation en outre l'organisation syndicale peut bénéficier d'une indemnité spécifique lorsque la collectivité territoriale lui retire le bénéfice d'un local mis à disposition pendant au moins 5 ans sans lui proposer un autre local, je vous remercie. Si la parole est à Madame soufi taillé pour Lyon pour répondre à Madame la secrétaire d'État. Merci madame la présidente, madame la ministre, effectivement vous le soulignez, les collectivités territoriales peuvent mais elles peuvent aussi décider du contraire et notamment de mettre fin à d'une occupation de locaux qui étaient pourtant pour les salariés et les organisations syndicales, alors effectivement c'est un demi adénite et sur 5 ans, mais après des organisations syndicales, c'est aussi le temps long et et la problématique ne sera pas résolu peuvent les collectivités effectivement peuvent le faire, mais elles peuvent aussi souhaiter d'arrêter pourquoi parce que elles sont toutes dans une situation qui est complexe, financièrement, elles ont certainement toutes besoin parfois de pouvoir retrouver la la le le le la, je dirais, l'usage d'un Patrimoine mis à disposition, il y a longtemps, je pense, et je crois que c'est très extrêmement important pour la liberté syndicale, la défense des salariés qu'il faut aller plus loin et aider les collectivités ou aider les les organisations syndicales à garder un pied dans dans ces territoires et ne pas leur retirer des moyens qui sont essentiels, notamment pour l'accès aux droits des des salariés qui n'ont pas pas la chance dans leur entreprise de d'avoir accès à ces organisations merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Mireille Jouve la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des Transports, la parole est à madame Mireille Jouve. Merci madame la présidente, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la saturation préoccupante de la gare Saint-Charles de Marseille pour y remédier, la réalisation d'une gare souterraine sous le plateau ferroviaire déjà existants, ainsi que la création d'une 4ème voie dans l'Est marseillais sont une impérieuse nécessité la remise en cause de ces projets d'aménagement porterait fortement atteinte au développement économique et urbain futur de la métropole Aix-Marseille-Provence, la montée en puissance des transports ferrés du quotidien au sein de cette terre et plus largement de l'ensemble des Bouches-du-Rhône représente une atteinte forte, une attente forte des usagers et des élus locaux devant l'importante saturation de nombreux axes routiers toutefois un report modal ambitieux ne saurait en s'envisager son 20 traitement du verrou que représente la gare Saint-Charles aussi alors que le gouvernement procède actuellement à une réévaluation de l'ensemble des grands projets d'infrastructures de transport en France, pouvez-vous me dire : Madame la Ministre, si la concrétisation du projet stratégique de traitement du noeud ferroviaire de la gare Marseille Saint-Charles demeure une priorité, je vous remercie. Merci de la parole est à madame brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre des tas, Ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous m'interpellez sur l'avenir de la ligne ferroviaire reliant moi. Vous m'interpellez sur le noeud ferroviaire de la gare de Marseille Saint-Charles, je tiens tout d'abord à vous affirmer le souhait du gouvernement d'améliorer le fonctionnement du noeud ferroviaire de Marseille et d'offrir aux usagers des liaisons régionales plus régulière et plus fiables sur l'ensemble de la ligne de Marseille à Nice, le projet de Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur a été conçu dans cet objectif-là, les études préalables à l'enquête publique, ont été menées et des approfondissements sont attendues s'agissant notamment des conditions de passage en tunnel dans la vallée de l'Huveaune néanmoins, comme vous le savez, le projet est très coûteux, les 2 sections prioritaire autour de Marseille et Nice étant estimé à près de 7 milliards d'euros dans un contexte où près de 35 milliards de projets financiers ferroviaires sont à financer dans l'ensemble de la France, c'est dans ce contexte que le gouvernement a mis en place une méthode particulière pour les grands projets d'infrastructures de transport avec les Assises de la mobilité qui sont menées depuis septembre et qui vont se clôturer prochainement la le 13 décembre et puis avec la loi d'orientation sur les mobilités début 2018, c'est une nouvelle politique de mobilité que nous souhaitons une politique qui soit plus à l'écoute des besoins de nos concitoyens mais aussi plus réaliste et surtout aussi plus sincères avec nos finances publiques, les débats sur ce projet, prendront toute leur part et toute leur place, il convient cependant de rechercher dès maintenant les optimisations possible des réseaux existants pour redonner rapidement de la régularité et de la capacité à nos services de transport noeud ferroviaire le noeud marseillais dont vous parlez, SNCF, réseau et mobilisés pour rechercher les moyens d'optimiser, non seulement les conditions d'accès au plateau de Saint-Charles, mais aussi les pratiques actuelles d'exploitation et les investissements pertinents à différents horizons 2024 d'abord, qui est la date des Jeux olympiques et par un olympique et puis en 2030 au-delà et même au-delà en fonction déphasage possible de la ligne nouvelle, ces réflexions, elles vont permettre d'éclairer les décisions qui seront prises dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités qui est à venir. Merci. Si la parole est à madame Mireille Jouve pourrait. Pondra madame la secrétaire d'État. Oui, je vous remercie de ces précisions, je voudrais rappeler que la métropole Aix- Marseille-Provence qui est en pleine construction, attend beaucoup de l'État, en particulier dans le domaine des transports, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet, mais je crois que les 92 communes qui la constituent, n'auront pas un budget suffisant pour ces grands projets, donc nous attendons vraiment beaucoup de l'État et puis vous avez bien fait de rappeler également que nous devons travailler l'art, l'accueil des Jeux olympiques qui verront certaines épreuves de voile se dérouler à Marseille, je vous remercie. ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des Transports, la parole est à monsieur Roland Courteau. Merci madame la présidente, 42 conseils municipaux de la haute vallée de l'aube, madame la secrétaire d'État et l'Association pour la ligne ferroviaire Carcassonne-Quillan, élus et population, décidé de s'opposer à la fermeture du tronçon ferroviaire Limoux, Quillan, si nous nous réjouissons de la régénération réalisé de la première partie de segments Carcassonne, Limoux, la menace de fermeture du 2ème segments Limoux, Quillan soulève la plus totale réprobation c'est ligne doit absolument rester un véritable outil de développement du territoire est un véritable levier économique, il ne sera pas accepté et je pèse bien mes non que la continuité ferroviaire Limoux, Quillan soit remise en cause, je porte à votre naissance, madame la secrétaire d'État au cas où vous l'ignore rien que la région a voté en juillet dernier, le financement de 610000 euros d'études étape constitutive à la réalisation des travaux et ces études je le précise, viennent de débuter, je rappelle que les populations considère que cette ligne doit rester dans le périmètre national afin de conserver en réseau garantissant l'unité, la continuité du territoire et l'égalité d'accès aux transports, il est donc demandé l'abrogation du décret portant sur les contrats de performances passées qui exclut les lignes de catégorie lycée cette à 9 de l'entretien et maintenance courant dans la ligne pré-cités je j'insiste d'ailleurs pour que SNCF raison mettent à niveau l'entretiennent de base afin de rétablir et garantir les performances de temps de parcours sur l'ensemble de la ligne, bref je veux rappeler ici, encore une fois l'engagement qui a été pris, ça la moindre ambiguïté par le conseil régional pour que soit inscrit des travaux de rénovation du tronçon Limoux, question madame la ministre, qu'en est-il des intentions du gouvernement et avec lui de la SNE SFR. Merci monsieur Courteau, la parole est à madame brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la présidente. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous m'interpellez sur l'avenir de la ligne ferroviaire reliant Carcassonne, Limoux et Quillan, dans l'auto, comme vous le savez l'état dégradé de cette infrastructure a conduit à la mise en place de limitation de vitesse sur plusieurs sections de l'axe pour maintenir un haut niveau de sécurité, la réalisation de travaux de renouvellement était dès lors nécessaire pour rétablir ce niveau de performance, les études menées dans le cadre du Super 2017 2007, 2013 ont permis de définir les besoins de régénération et les travaux à effectuer en priorité pour assurer la pérennité de cette ligne, l'État et la région ont ainsi validé une enveloppe de 11 millions d'euros, actant un engagement fort pour traiter la section entre Carcassonne et Limoux, où circule le plus grand nombre de trains, les travaux les travaux ont commencé depuis début 2017 et ils vont se poursuivre encore en 2018, la section Limoux, Quillan présente quant à elle, en plus d'un état de vieillissement qui est avancé une configuration géographique complexe et qui impose des mesures garantissant la sécurité de circulation à ce stade et dans un contexte budgétaire qui contraint pour l'ensemble des acteurs d'ailleurs la priorité donnée aux partis structurants du réseau ne permettent pas à SNCF, réseau d'investir seul dans la pérennisation du réseau secondaire ni à l'État d'y consacrer en priorité c'est moyens l'avenir de ces lignes peut circuler comme Carcassonne-Quillan ne peut donc se construire qu'en partenariat avec la région et dans le cadre du CPE Les états généraux du rail et de l'Inter Mohamed mobilité qui sont organisées par la région Occitanie sont allés dans ce sens, ils ont d'ailleurs permis de définir les priorités en terme de mobilité durable à l'échelle régionale, il a été décidé de rechercher le maintien de la ligne dans tout son linéaire, une étude préliminaire de ligne sur la section Limoux, Quillan va ainsi être lancée rapidement, pour déterminer les conditions de ce maintien de services. Parole est à monsieur vous ne souhaitez pas répondre à madame. La secrétaire d'État, je vous remercie, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Jean-François Longeau au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, la parole est à monsieur Longeau. Longeau. La présidente, madame la ministre ma question après sur la baisse annoncée dès budget des agences de l'eau depuis la loi de finances 2015, l'État en plus chaque année, le fonds de roulement des agences de l'eau de près de 175 millions d'euros pour financer son propre budget, sans compter une diminution drastique et imposer des effectifs ces prélèvements se font détriment des collectivités, bien entendu et missions des agences de l'eau sans cesse élargi sans cesse renforcés à l'heure où l'État demande aux collectivités drogue anisée les compétences, eau et assainissement sur leur territoire et de mettre en oeuvre la compétence j'aime Mappy cette diminution prévue des Budgets des agences de l'eau, si elle est entérinée, mettrait à mal les investissements prévus par les collectivités locales pour accompagner la transition écologique, effectivement, il y a de nombreux dossiers de mise aux normes, à la fois des réseaux, des stations d'épuration et nombreuses sont les maires qui se pose la question de savoir comment ils vont pouvoir financer ces travaux Madame Émilie, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'indiquer si il est dans vos intentions dans les intentions du gouvernement de préserver l'autonomie financière et administrative des agences de l'eau, je vous remercie. Merci, la parole est à madame brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la présidente. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous interrogez le ministre d'État de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, il ne peut malheureusement pas être présent aujourd'hui et c'est pour ça qu'il m'a chargé de vous répondre depuis sa prise de fonction, Nicolas Hulot a rencontré à 2 reprises l'ensemble des présidents de comités de bassins et des directeurs des agences de l'eau, la conviction du ministre d'État et que leur gouvernance par bassin a du sens et que ce type de gouvernance là doit être respecté et préservé les agences constitue un fantastique outil au service des politiques de l'eau mais également de la biodiversité de l'adaptation au changement climatique, cela dit, il nous semble néanmoins que certaines évolutions sont devenues nécessaires d'abord, les agences de l'eau doivent avoir un rôle de pilier dans le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité, c'est bien dans ces tests dans cet esprit-là qu'vont désormais financer entièrement les opérateurs de la biodiversité, l'Agence française de pour la biodiversité, les parcs nationaux et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pourquoi, parce que le lien est évident entre la gestion de l'eau et la gestion des écosystèmes. S'agissant des moyens, des agences de l'eau, ceux-ci sont et restent très importants ainsi au-dessus du 11ème programme nous prévoyons plus de 12,6 milliards d'euros de recettes fiscales sur 6 ans, cette somme est exactement intermédiaire par rapport aux 2 programmes précédents qui s'était vu allouer 13,6 milliards d'euros et pour le 10ème programme et 11,4 milliards d'euros pour le 9ème programme pour l'année 2018 les plafonds des redevances qui pourront être collectées au profit des agences de l'eau devait être abaissée, il a été remonté à 2,28 milliards d'euros à la demande des députés en contrepartie de cette hausse du plafond Le gouvernement réintroduit un prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau à hauteur de 200 millions d'euros, ces 200 millions d'euros, là ils sont destinés à les comparer au fonds de roulement qui s'élevait à 760 millions d'euros fin 2016 et ils correspondent environ à la hausse de ce fonds de roulement entre 2014 et 2016 malgré les prélèvements opérés sur cette période, par ailleurs, nous avons un enjeu majeur autour de l'amélioration de l'état des réseaux d'eau et de la gestion de ces réseaux d'là, c'est pourquoi le président de la République a annoncé à l'occasion du congrès des maires, la tenue d'Assises de l'eau, ces assises, elles vont être lancées par le ministre d'État, l'année prochaine, elles vont permettre de regarder finalement en détail avec granularité les besoins d'investissement qui concernent ces réseaux-là, on le sait, ils sont importants, sachez en tout cas que nous veillerons à permettre à chacune de ses agences ont découvert, madame la maire d'exercer pleinement leur mission dans le cadre de ce 11ème programme cette priorité partagée par les présidents de comités de bassin. Merci, la parole est à monsieur longs jours pour répondre à Madame la secrétaire d'État. Oui merci madame la Miss, moi j'ai bien entendu effectivement qui avait des évolutions nécessaires et et participera à ses évolutions nécessaires qu'il faut mais simplement quand même si on veut bien entendu mettre en rien à la gestion de l'eau et des écosystèmes, il faut quand même et c'est logique, mais il faut quand même qu'il y a des moyens et je crois qu'aujourd'hui notre difficulté dans la gestion des collectivités, c'est, c'est un véritable manque de moyens dans le domaine de de l'eau et l'assainissement et que bien sûr, si les enjeux majeurs sur les réseaux d'eau, feront l'objet d'assise et autres, je crois que c'est important, parce que je crois que notre avenir passe par la gestion de l'eau aussi des des je crois que c'est des dossiers très importants, mais je crois qu'il faut dans ce domaine, faire confiance aux collectivités qui ont géré l'eau jusqu'à maintenant d'une façon remarquable mais leur faire confiance aussi, c'est essayer de leur donner des moyens et c'est ce que je souhaite, dans les années à venir, et j'espère que ces assises nous permettra de trouver des moyens de, de, d'accompagner les collectivités locales et puis de se rappeler quand même quelque chose mais ce n'est pas uniquement pour ce gouvernement puisque ça fait des années qu'il y a des et des prélèvements sur les agences de l'eau mais que normalement la redevance payée par les sur les factures d'eau concerne effectivement l'eau, il ne doit pas être dans un budget, quel qu'il soit, merci.

dans un rapport consacré à la gestion des enseignants, la Cour des comptes, a déploré le caractère imprévisible et lisible de la politique de recrutement de l'État, les gouvernements précédents ont mis en 9 des mesures manquant de cohérence au regard de la nécessaire stabilité à long terme de l'Éducation nationale, ainsi les effectifs des enseignants et la démographie des élèves ont évolué différemment, en particulier dans le second degré, comme le souligne la Cour pour les étudiants, envisageant d'exercer ce métier ces incohérences ont eu un effet dissuasif incontestable, le taux de candidats présents au concours néant cessé de diminuer entre 2012 et 2015 en outre tous les postes ouverts n'ont pas été pourvu que ce soit dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire, ce qui a eu pour effet d'aggraver la situation dans un certain nombre d'établissements, mais le manque d'être il d'attractivité du métier d'enseignant a aussi des causes plus profondes, la faiblesse des rémunérations en début de carrière, l'insuffisance de la formation professionnelle continue et l'imparfaite, procédure d'affectation des enseignants incite fréquemment les jeunes à se tourner vers le secteur marchand qui offrent de meilleures perspectives de carrières et des rémunérations plus attrayantes, les conséquences sont lourds pour les établissements scolaires toutes les filières, la filière générale, la filière technologique et la voie professionnelle sont affectés par la faible capacité de séduction de l'Éducation nationale, certaines disciplines comme les sciences et les mathématiques connaissent de réelles difficultés de recrutement, et il est parfois nécessaire de recourir à des enseignants contractuels pour assurer la continuité des cours et faire face à un absentéisme qui pénalise les élèves dans mon département, l'Essonne, il manque des enseignants spécialisés dans certains établissements, j'en veux pour preuve la situation du lycée de l'essor You aux Ulis qui a recherché jusqu'aux vacances de la Toussaint, des profils très technologique, cette situation est évidemment très dommageable pour des élèves qui préparent l'orientation professionnelle future, donc ma question sera précise, Monsieur le Ministre, si les premières mesures prises par le gouvernement semble aller dans le bon sens comment comptez-vous faire face aux défis du recrutement des enseignants et donner à nos enfants les moyens de réussir leur scolarité et leur insertion professionnelle, je vous en remercie. Merci, la parole est à monsieur Jean Michel Blanc Ministre de l'Éducation nationale. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice par Darcos c'est une question évidemment importante, c'est même la question cruciale de tout système éducatif et il y a plusieurs questions dans dans votre question, d'abord, on doit faire une distinction entre le 1er degré et le second degré, la crise dont vous parlez est fondamentalement une crise du second degré dans le 1er degré les 13000 postes proposés aux concours et qui vont continuer à être de cet ordre de grandeur avec les créations de postes que nous faisons dans dans le 1er degré sont pourvus, on pourrait discuter de l'attractivité de la fonction de professeur des écoles, mais elle ne connaît pas une crise trop grave en revanche dans le second degré, nous avons une crise importante y a une dimension mondiale et puis une dimension française la dimension mondiale, c'est que, on observe que certaines disciplines manque d'attractivité pour la fonction professoral, c'est particulièrement vrai pour les mathématiques et disciplines scientifiques et technologiques comme comme vous venez de le dire, ce phénomène on doit donc le on va voir la dimension structurelle et le contre-et puis il y a des dimensions peut-être proprement française qui sont liés peut-être avait effectivement au problème de gestion que vous avez mentionné sur la dimension la plus importante, la plus structurelle, là il y a évidemment une série de réponses, mais la première d'entre elles, la plus importante, c'est le pré-recrutement, nous devons être capables au cours des prochaines années d'inciter des jeunes qui ont des dons ou de ou et des désirs de carrière en mathématiques, en sciences en technologie à se diriger vers ces carrières et de façon plus générale l'dans l'ensemble des disciplines, on doit inciter à cela, on doit le faire avec des mesures matérielles et immatérielles sur le plan immatériel, c'est peut-être le plus important c'est la valorisation dans notre société de la fonction de professeur, c'est ce que je fais tous les jours et que je vais faire encore maintenant en répondant sur la question de ce que nous dit l'enquête Pearl, le professeur doit être au centre de la société française, il doit être valorisé dans tous les sens du terme, et puis, d'un point de vue plus pratique, ce sont les bourses que nous allons développer en matière de de pré-recrutement, ce sont aussi, c'est aussi l'évolution de la fonction d'assistant d'éducation qui va nous permet de diriger plus d'élèves et d'étudiants vers la fonction professoral dans le futur, cela se doit se traduire par plus de candidats au concours, nous devons être aussi attentif à la qualité de ceux des concours puisque dans le passé trop souvent la barre d'admission, a été mise bas et même en la mettant bas, les concours n'ont pas été pourvus, parfois avec des taux de 85 pourcent, en moyenne, mais ça va peut descendre plus bas pour les disciplines que j'ai évoquais donc il faut recréer de l'attractivité, le faire progressivement rehaussé la barre de de l'exigence, c'est le cercle vertueux de la qualité du système français qui est en jeu et c'est ce que nous avons commencé à engager merci beaucoup. Merci monsieur le ministre, la parole est à madame Lord Arcos pour répondre à monsieur le maire. enfin, bien évidemment, de tout coeur avec vous, je pense que la représentation nationale et et derrière vous dans, dans, dans ses travaux et j'espère que vous pourrez rester 5 ans ministre de l'Éducation ational parce que je pense qu'il faut au moins 5 ans pour que vous puissiez peut-être mener à bien vos réformes, merci monsieur ministre. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Pierre Ouzoulias au ministre de l'Éducation nationale la parole est à monsieur Ouzoulias. merci madame la présidente, monsieur le le ministre votre ministère utilise beaucoup de critères d'indicateurs pour pour classer les établissements notamment, et c'est comme ça que vous déterminer quels sont les établissements qui doivent appartenir au réseau d'enseignement prioritaire et au réseau d'enseignement prioritaire plus ces critères, sachez-le, sont aussi utilisés par les collectivités, je pense notamment au département pour ajuster les moyens qu'il donne aux établissements en fonction de, de vos de vos classement, donc ils ont une une double utilité qui qui parfois provoque des effets de levier qui sont, qui sont importants, sur le terrain, il nous semble parfois que l'évolution du classement des établissements ne correspond pas tout à fait à la réalité sociologique du terrain, telle que nous la percevons nous c'est évidemment un un critère très subjectif dans mon département, Les Hauts de Seine, j'ai demandé à plusieurs reprises qu'on me communique ses critères pour essayer de comprendre le le décalage entre ces cette quantification est ce que je percevais et on m'a dit que ce n'était pas possible, c'était des critères qui étaient propres ministère et que je n'avais pas il y accéder sur le fond, je trouve que c'est pas, c'est plus une façon acceptable aujourd'hui de faire de la bonne administration et je crois que vous savez Monsieur le Ministre, ce que je pense que sur ce point-là on on partage la même opinion que pour les critères, comme pour les algorithmes, la seule façon de bien les protéger, c'est la rende publique et d'en discuter de façon politique, donc ça c'était ma première question, quand est-ce qu'on pourra obtenir la publication de ces critères, la seconde, et vous me voyez venir parce que on a eu une discussion là-dessus lors de la discussion du budget, c'est : quid de l'extension de ces critères aux établissements privés sous contrat, parce que là aussi on a besoin d'évaluer, nous en tant que politique qui subventionnons ces établissements, quelle est leur part dans la lutte contre le le décrochage scolaire qui passe aussi par une une meilleure mixité sociale au sein des des ADP des établissements Jean merci. merci. Si la parole est à monsieur Jean Michel Blanc Ministre de l'Éducation nationale. pour cette question qui est elle aussi très importante et qui porte sur l'éducation prioritaire, qui est sujet essentiel pour pour pour notre pays, il y a donc 2 volets : la 1ère sur les critères de de l'éducation prioritaire, il est exact que l'éducation nationale depuis la création même du concept au au début des années 80 a développé un savoir-faire sur la définition de ces critères et que le le résultat auquel on arrive, et dans l'ensemble assez satisfaisant, même si ça n'est pas, je vous l'accorde volontiers pleinement satisfaisant, je suis totalement d'accord avec vous sur l'enjeu de transparence des algorithmes et de transparence des critères et donc nous allons nous diriger vers cela dans peu de temps et Jacques céderait volontiers à ce que vous dites, d'autant plus que nous devons viser une cohérence entre les politiques publiques de l'éducation prioritaire, et les politiques publiques, sociales de façon générale et que nous, de la direction que nous devons prendre, c'est aussi de faire de l'établissement, souvent, le pivot des politiques sociales, je pense à tout ce qui a trait, notamment, relations avec les familles, à l'aide aux familles à l'aide à la parentalité qui est évidemment intimement lié à ce qui se passe dans le 1er degré dans le second degré dans les territoires les plus défavorisés, donc en lien avec la représentation nationale, nous pouvons tout à fait progresser en en la matière, nous devons progresser sur notre conception de l'éducation prioritaire, qui certes à une dimension territoriale mais en réalité, nous avons des élèves défavorisés aussi en dehors des territoires définis comme étant de l'éducation prioritaire, et doit donc y avoir à la fois une approche sociale territoriale à une approche sociale plus plus individualisé, c'est aussi le sens d'évolution que l'on vous proposera dans les dans les dans les prochains temps mais là aussi j'adhère à à l'esprit de votre de votre question, ensuite le sur le la 2ème partie de votre question qui est l'application de la notion d'éducation prioritaire à l'enseignement privé, je trouve que c'est un point très intéressant parce que, en effet, il y a une participation réelle et volontariste de l'enseignement privé sous contrat aux enjeux de mixité sociale, mais cette participation n'est pas la même selon les les les lieux que l'on considère en France et même, selon d'autres critères que les territoires, on devrait, on doit donc être attentif à cette question et c'est aussi une évolution, je discuterai évidemment avec les partenaires sociaux et avec les partenaires de de l'enseignement privé, mais ça me semble être une remarque qui va dans la dans la bonne direction, puisqu'il y a de la volonté de la part de l'État mais aussi des acteurs concernés, de jouer un rôle plus important dans le domaine de la mixité sociale et et de et du travail en faveur des élèves les plus défavorisés socialement. Merci monsieur le ministre, la parole est à monsieur Ouzoulias s'pour répondre à monsieur le ministre. Merci monsieur minutes pour vos réponses claires et et honnête je voulais juste rajouter un petit point sur la constitution des critères de détermination des rangs sociaux des des des établissements, il nous semble, à l'usage que il est fait une une grande part au système déclaratif, c'est-à-dire qu'on demande aux familles de déclarer leur situation sociale, or il se trouve que c'est dans les établissements les plus défavorisés que les parents remplissent le moins cette cette situation, un effet un peu un peu particulier et qui est et qui a tendance à faire que, malheureusement, c'est dans les secteurs les plus que les critères sont les moins efficaces, ce qui est ce qu'un souci, par ailleurs, votre volonté que je partage pleinement, d'essayer de restaurer un peu de mixité sociale dans les établissements en région parisienne, elle se heurte à une ségrégation territoriale dont vous n'êtes pas responsable mais donc, mais donc vous avez malheureusement à gérer les effets, c'est-à-dire que, pour reprendre le département d'que je connais aujourd'hui la ségrégation territoriale qui a chassé une une bonne partie des des familles pauvres vers uniquement à 4 ou 5 territoires fait que, à l'échelle d'une commune, il y a plus de possibilité de mixité sociale, tout à fait tout, c'est tout à fait dramatique Jean merci. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Hélène Conway Mouret à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, la parole est à Madame Conway mourez. Merci madame la présidente, madame la ministre mais, chers collègues, cette question orale s'inscrit dans le prolongement d'une question écrite que j'ai posée au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a quelques mois, je souhaite attirer l'attention de l'ensemble des administrations impliquées dans l'accueil des étudiants français venant de l'étranger dans la procédure de demande de bourse et de logements universitaires gagnerait à être modernisé et simplifier un constat tout d'abord un certain nombres d'étudiants viennent seulement de recevoir au mois de novembre 2017 une notification relatives à leur demande de bourse universitaire pour l'année en cours alors qu'ils en avaient fait la demande dans les délais, cela s'explique par les lenteurs de transmission de leur dossier social étudiant entre leur pays de résidence et la France, il rate de la même façon, les tours d'attribution de logements dans le parc universitaire, c'est évidemment une grande injustice pour eux et pour leurs familles qui doivent avancer les frais d'inscription de Sécurité sociale et trouver des logements dans le parc privé, avec les difficultés que l'on connaît, je ne rentrerai pas ici dans le détail du circuit de transmission de ce dossier qui va du demandeur ocre ou s'en passant par le consulat, le tout en partie par voie postale dans des pays où la Poste n'est d'ailleurs pas toujours très fiables, mais il est évident que la dématérialisation de cette procédure, constituerait un gain de temps pour tous, j'aimerais donc savoir si vos services, madame la ministre, il travaille le formulaire de demande de bourse et de logements universitaires en lui-même est calqué sur celui des bourses scolaires, il est donc pas adaptée en l'état actuel du barème d'attribution des bourses, 2 points de charge sont accordées aussi bien un jeune Français qui arriveraient seuls d'Amérique du Sud, qu'un jeune Lyonnais quitterait Lyon pour s'installer à Lille a minima le bonus accordé sous forme de points de charge aux jeunes partant faire des études à plus de 250 km du domicile familial devait très devrait être majoré pour les futurs étudiants qui arrivent de l'étranger, plus largement, il conviendrait d'appliquer des points de charge en concordance avec le vécu de nos compatriotes à l'étranger qui supporte des frais élevés de scolarité et d'assurance maladie, enfin concernant les logements, j'aimerais savoir s'il serait possible d'accorder à niveau de bourse équivalent la même priorité aux étudiants français qui viennent de l'étranger aux ultramarins dont les contraintes sont similaires, je vous remercie, Madame la Ministre, de vos précisions sur les améliorations que vous pourrez apporter au système avant la prochaine campagne. Merci, la parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Hélène Conway Mouret mais jamais sénatrice, messieurs les sénateurs, vous attirer mon attention sur la situation des étudiants français vivant à l'étranger, au regard de leur demande de débourser de logements en résidence universitaire, comme vous le savez, l'amélioration des conditions de vie des étudiants pour favoriser la réussite tout au long de leur parcours, constitue l'une des priorités de l'action gouvernementale et j'y reviendrai, la définition des modalités d'attribution de bourses universitaires aux étudiants français de l'étranger, repose sur une circulaire rédigée par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle relevant de mon ministère, il est donc tout à fait possible que nous puissions travailler sur cette circulaire, qui prend en compte le niveau de vie des parents à travers leur situation familiale et leurs revenus et prend en compte aussi l'éloignement entre le domicile de la famille est le lieu d'études, même si, comme vous l'indiquez, les choses sont probablement perfectible sur ce sujet puisque la limite est ici est une attention particulière et de surcroît porté aux étudiants qui font le choix d'étudier, loin de leur territoire d'origine et je pense aux étudiants, visés par votre question, mais aussi à nos compatriotes ultramarins qui effectivement bénéficient de conditions qui peuvent être différentes et qui pourraient être harmonisés en tout cas un travail en ce sens, peut effectivement être être à moyen terme, plusieurs mesures qui sont mises en avant dans le cadre du plan étudiant j'ai présenté le 30 octobre dernier permettront de réduire le coût de la rentrée pourront au moins partiellement, répondre à vos questions dès 2018, plus aucun étudiant ne cotisera à une à un régime de Sécurité sociale spécifique et tous les étudiants seront rattachés au régime général de la Sécurité sociale, la simplification du circuit de traitement des bourses a été ouvert avec les ainsi que celui d'une aide globale d'autonomie qui fait l'objet d'une réflexion approfondie, actuellement à la fois auprès des services du ministère mais aussi plus généralement avec les collectivités, l'opportunité d'une aide spécifique à la mobilité apprécier au cas par cas, est également à l'étude, notamment dans le cadre de l'ouverture des quotas de mobilité inter-académiques, présenté dans le projet de loi d'orientation et de réussite des étudiants que vous aurez à voir très rapidement concernant les logements étudiants, nous espérons aussi que la construction de 60000 nouveaux logements réservés aux étudiants permettra de répondre à cette épineux problème merci.

il ne recherche pas un passe droit ou un privilège pour ces jeunes bacheliers français qui ont passé leur bac à l'étranger mais aujourd'hui un peu dommage que ceci alors que souvent ils ont de très bons résultats avec un un taux de de mentions très élevé que pour des blocages administratifs, il ne puisse pas continuer leurs études et les faire en France et qu'soient forcés, aller dans un autre pays que le mien que lui, que le nôtre, pardon et soit forcés d'étudier ailleurs, je note avec satisfaction votre volonté d'apporter un peu d'égalité dans un système qui en fait aujourd'hui est discriminatoire et qui est est ressentie par beaucoup de familles comme une injustice, alors que les règles peuvent être assez facilement changer simplifier la dématérialisation permettrait je pense, de faire en sorte que les demandes qui viennent de l'étranger soit faite dans les délais, parce qu'il il les respecte mais malheureusement à cause de la Poste, leur demande arrive toujours trop tard, donc je vous remercie pour tout ce que vos services pourront mettre en place pour aider toutes ces familles et ces jeunes merci. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Alain jouions d'être transmise au ministre de la cohésion des territoires, la parole est à monsieur Merci madame la présidente, monsieur le ministre, d'abord merci de votre présence, le projet de loi de finances pour 2018 est actuellement en débat au sein de notre assemblée contient plusieurs mesures fiscales relatives au logement, qui sont de nature à susciter de l'inquiétude, tant pour les classes moyennes et les territoires ruraux que pour l'emploi, la première mesure qui est prévue à l'article 40 consiste à recentrer le prêt à taux 0 pour les constructions neuves dans les secteurs immobilier plus en tension. Or, l'exclusion des zones les moins tendue, constitué principalement de territoires ruraux aura pour effet d'exclure de ce dispositif, les populations qui vivent alors qu'elles ont bénéficié, actuellement le plus parallèlement le recentrage du prêt à taux 0 pour les logements anciens dans les secteurs immobilier l'est moins en tension, cette fois-ci, n'est pas plus acceptable conjugué au recentrage du prêt à taux 0 pour les constructions neuves, il restitue une ségrégation entre les candidats à l'accès à la propriété, selon le territoire où il souhaite s'établir. Avec ses premières mesures, on peut désormais dire aux territoires urbains des logements neufs et aux territoires ruraux des logements anciens, deuxièmement, de la même manière, la 2ème, mesure prévue à l'article 39 s'inscrit totalement dans la philosophie de la première, elle procède au recentrage de la loi dite Pinel au même zone tendue, ce qui aura pour effet de concentrer encore plus les investissements immobiliers locatifs dans les territoires urbains, voire très urbain, la prorogation des prêts à taux 0, la loi Pinel au 31 décembre du 31 décembre 2017 2021 prévue par le projet de loi de finances va dans le bon sens, néanmoins le recentrage globale en direction des zones et plusieurs aura pour effet d'accentuer un peu plus la fracture territoriale de notre pays, et davantage encore la politique d'aménagement du territoire de la République en concentrant la politique fiscale relative aux investissements immobiliers résidentiels ou locatif dans quelques grandes villes, on y concentrera inévitablement les populations et l'activité économique, alors qu'il faudrait plutôt orientées les politiques publiques en faveur du développement des territoires qui sont naturellement les moins dynamiques, la 3ème mesure consiste à remplacer l'actuel crédit d'impôt pour la transition énergétique par une prime éponyme à partir de 2019, cette mesure, si elle n'est pas prévu en tant que tels, par le projet de loi de finances 2018 est anticipé entre autres par la sortie des chaudières à fioul et des menuiseries du crédit d'impôt pour la transition énergétique d'ici le 30 juin 2018, monsieur le ministre, toutes ces mesures ajoutées inquiète terriblement nos territoires évidemment je suis impatient de la réponse que vous allez me faire. Merci, la parole est à monsieur Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Merci madame la présidente, monsieur le ministre Joyandet, je crois que votre question qui est certes tout à fait pertinent qui ne correspond pas tout à fait à la réalité de ce que nous sommes en train de faire d'abord parce que en ce qui concerne le prêt à nous allons aboutir à une solution qui me paraît au contraire parfaitement équilibré puisque ce prêt à taux 0 est maintenu, vous savez que, que ce soit loi Pinel au prêt à taux 0, cela devait s'arrêter le 31 décembre 2017, le gouvernement a pris la décision de prolonger le dispositif Pinel pour 4 années dans les secteurs tendus et en ce qui concerne le prêt à taux 0, il y aura bien évidemment en ce qui concerne les territoires dits détendus, 4 ans pour l'ancien, et 2 ans pour le 9, donc nous avons non seulement prolongé de plus d'une année pour donner de la visibilité de la visibilité aux constructeurs et à ceux qui veulent investir dans le logement en ce qui concerne en outre la question du CICE nous envisageons pour 2019, de mettre en place une prime, qui sera pour chaque Français qui voudra investir dans ce secteur, en plus, beaucoup plus une solution beaucoup plus simple à utiliser et puis il faut pas faire, je crois, un procès au gouvernement par de laisser de côté les territoires ruraux ou les classes moyennes, dans la mesure où je suis en train de mettre en place un plan spécifique pour les villes moyennes, ce qui n'avait pas été fait depuis. Beaucoup de décennies pratiquement depuis les années 1970 et je crois que, à ce niveau-là, au contraire, c'est un dispositif qui permettra de rétablir un équilibre qui avait été pour le moins fragilisé avec la métropolisation que nous connaissons, qui est certes utile mais qui avait laissé un peu de côté nombres de villes moyennes, donc j'ai signé récemment un protocole d'accord avec Action Logement qui investira un milliard et demi sur les villes moyennes dans les 5 ans, le gouvernement va remette de l'ingénierie mettre une série de dispositifs aussi en coordination avec la Caisse des dépôts sur ces villes moyennes qui irrigue les territoires ruraux qui sont autour, donc cette préoccupation, c'est la nôtre, monsieur le ministre et nous allons faire en sorte d'aller je pense dans ce sens-là, qui correspond à votre objectif. Merci monsieur le ministre de la parole est à monsieur Alain Joly, un téléfilm répondre à Monsieur le Ministre. Merci la la présidente, merci monsieur Ministre pour votre votre pour avoir siégé avec vue sur ses bancs, je sais que vous êtes sensible à l'équilibre dès l'équilibre des territoires je pas toujours facile pour vous de gérer les textes actuels, j'ai bien compris que, du coup, vous aviez de nouveaux projets pour contrebalancer, donc je vous en remercie, mais pour l'instant, l'état du droit, cette ces nouvelles intentions sont encore une attente pour nous et nous verrons quand, quand tout ça viendra simplement je veux vraiment insister sur cette inquiétude qu'on a dans nos territoires, parce que souvent c'est la double peine, c'est la double peine pour nos territoires, puis c'est la double peine aussi pour les classes moyennes, parce que souvent, ces classes moyennes habitent nos territoires et donc voilà, je voulais vous faire part ce matin de cette inquiétude qui est ressentie par nos élus locaux par les classes moyennes qui vivent dans nos territoires ruraux, merci pour cette annonce concernant les villes concernant les villes moyennes, mais je pense qu'il faut vraiment rester très très attentif parce que, derrière, nous avons aussi derrière toutes ces mesures, les professionnels du bâtiment qui sont un peu inquiets, il y a de quoi donc merci pour les nouvelles annonces et nous attendrons, bien entendu, ces nouveaux travaux parlementaires, j'imagine, qui viendront dans les, dans les mois qui viennent et nous serons évidemment à vos côtés pour vous aider dans toutes ces dans tous ses objectifs partagés d'un bon équilibre de nos territoires, pour une meilleure vie pour tous nos concitoyens qui ont fait le pari d'y vivre avec leurs enfants, merci Monsieur le Ministre. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Pascal Savoldelli, au ministre de la cohésion des territoires, la parole est à monsieur Savoldelli. Madame la présidente, monsieur le Ministre, Madame la Ministre aussi et puis, mes chers collègues, donc le préfet de la région France doit avoir remis maintenant au 1er ministre les conclusions de la consultation opérer auprès des élus locaux et des différents acteurs qui font la métropole d'aujourd'hui évidemment. Les conclusions revient à l'exécutif national. Pas de sujet de ma part, par contre, quelles dispositions sont prises pour que la consultation soit rendue publique. C'est-à-dire restituer aux élus locaux. C'est-à-dire restituer à la population, nous savons qu'il n'y a pas consensus, d'abord parce que le cas de cette consultation est flou, il est franc, car l'initiative vient d'en haut et non pas des élus locaux, ni même à ma connaissance, d'une forte volonté de l'opinion publique mais un constat est partagé : oui, la métropole n'est pas à la hauteur des problèmes que rencontrent les habitantes et les habitants d'Île-de-France dans leur vie quotidienne, je me permettrai 2 exemples, il y a encore 640000 demandeurs de logement chaque année pour seulement 80000 attributions Jean prendre un second des autorisations d'installation des bureaux entreprises se concentrent à la Défense et dans l'ouest de la capitale et crée un déséquilibre économique profond dans le même temps, le triptyque, communes, départements, régions et dynamique. Et je m'attarder particulièrement sur l'échelon départemental, petite couronne comme grande couronne la l'action des départements leur leur appui aux communes leurs services publics de proximité, de solidarité sont très appréciés, Terres appartement permet des avancées qui profitent à toute la métropole, je pense au 1er tramway le T1, c'était un projet du département de la Seine-Saint-Denis mais je pourrais parler du 1er métro de banlieue à banlieue, la future ligne 15 Sud il reprend le tracé d'Orbival lancée par le département du Val-de-Marne, si les habitants, élus et agents territoriaux sont inquiets, c'est avant tout pour l'avenir, ces politiques-là et je pense que la déclaration du président de la République qui stipule en juillet dernier, vouloir, je le cite : supprimer 2 échelons en-dessous de l'échelon régional, monsieur le ministre, je dirais que quand il y a un flou, il y a souvent un loup alors qu'en est-il aujourd'hui au regard de tous ces éléments, pouvez-vous nous mais piquer en quoi les départements seraient un obstacle à la construction métropolitaine, merci pour votre réponse. Merci, la parole est à monsieur monsieur Jacques Mézard, ministre de la cohésion des terrils. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, je ne vais pas vous donner une réponse à une question qui n'est pas tranché. Vous nous dites : finalement le système aujourd'hui ne fonctionne pas bien et vous avez pris 2 exemples pertinents, mais ça va pas mais faut rien changer, ça c'est pas possible, si le président de la République a pris l'initiative de s'exprimer sur la question du Grand Paris, c'est que nous savons tous ce qu'il y a un problème que la situation actuelle : le fonctionnement actuel est extrêmement compliquée, si vous nous dites, nos concitoyens ne s'en émeuvent pas, moi je peux vous dire et vous le savez aussi bien si ce n'est mieux que moi que la complexité du système actuel, c'est que personne n'y comprend rien au niveau de nos concitoyens parce que il y a un réel problème sur l'articulation générale qu'est-ce que nous faisons, nous consultons effectivement que ce soit au niveau du du préfet de région, que ce soit à mon niveau, que ce soit au niveau du du 1er ministre moi j'ai personnellement reçu pratiquement toutes les associations d'élus toute la représentation des collectivités locales, donc je retire un élément clair c'est que tout le monde me dit le système actuel n'est pas bon ensuite, quant aux propositions qui émanent des différents de la représentation des collectivités c'est. le système actuel n'est pas bon, mais en ce qui concerne notre strate, ça fonctionne très bien, allez-vous donc voir sur telle autre strate si il ne serait pas bon de les supprimer, je résume, non pas de manière caricaturale et vous savez aussi bien que moi, Monsieur le Sénateur que ça c'est transcourant au niveau des sensibilités parce que là on est pas dans un affrontement droite-gauche, centre actuelle majorité l'histoire l'historique de ce qui s'est passé sur l'arrêt sur l'Île-de-France fait que on en est arrivé dans cette situation donc consultation effectivement tout le monde s'est exprimé tout le monde a pu s'exprimer tout le monde continue à s'exprimer et le préfet de région Île-de-France est travaille aujourd'hui pour faire la synthèse de de ses consultations d'un certain nombre de propositions, bien sûr, ce n'est pas encore tranché, ce que la consultation est en cours, vous nous dites : les départements vont être supprimés. Pour moi, ce n'est pas aujourd'hui actée, parce que nous sommes toujours dans cette réflexion, bien sûr il faudra améliorer le système actuel, nous en sommes tous conscients et c'est ce à quoi nous travaille. Merci monsieur le ministre de la parole est à monsieur Savoldelli pour répondre à Monsieur le Ministre. Monsieur le ministre, j'entends bien la difficulté de répondre. Ce qui manque déjà prononcée, quelle est l'ambition démocratique, sociale, économique de cette réforme territoriale de l'agglomération parisienne, Donc quand on la réclame ça veut-on dire qu'on est pas dans le statu quo, personne ne cherche l'immobilisme mais il faut bien qu'on propose à nos populations un projet donc là je vois qu'il y a une difficulté, je je ne vous la Mais c'est pour ça que quand je dis y a du flou, il y a un loup c'est quelle est l'ambition démocratique, sociale, économique pour l'Inter agglomération parisienne la 2ème chose c'est la question des consultations, vous savez tous, on est tous conscient qu'il y a une crise de légitimité de la politique, ça touche aussi les élus locaux, donc je pense que quand le gouvernement, l'exécutif national consulte les élus locaux, il revient à eux-mêmes, d'exprimer leur point de vue et vous avez raison, il y a une diversité de de points de vue mais il est du rôle du gouvernement de rendre à la population, cette consultation peut pas, elles doivent la fois faire l'objet d'une synthèse mais elles doivent être restitués aux populations, donc moi je le redis ici je suis nous sommes favorables à ce que la consultation des élus de toutes sensibilités, quelles que soient les niveaux maire président département la présidente de la région soit rendu pour que les citoyens se se fassent leur avis sur ce qui va évoluer la d'un chose que je veux dire c'est que nous, dans le Val-de-Marne, excusez-moi, mais 75 pourcent des des Val-de-Marnais, un sondage IFOP eux répondent, qui sont opposés à la suppression des départements et 71 pourcent demandent une consultation pas référendum donc il y a une aspiration des citoyens à avoir conscience de qu'est-ce qui va se passer du point de vue de leur quotidien, que vont devenir les services publics. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Jean-Louis Masson au ministre d'État, ministre de l'Intérieur Monsieur Masson, là vous avez la parole. Oui, mais question donc s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et je voudrais rappeler que le gouvernement et le président de la République, ont annoncé qu'il y aurait un certain nombre de réformes électorales et j'aimerais obtenir plusieurs précisions tout d'abord, pour ce qui est des députés et des sénateurs, je souhaiterais connaître une orientation du calendrier de la réforme, c'est-à-dire quand ce qui va être présenté au Parlement et savoir si la réduction fin du de la durée des mandats dans le temps, fera partie de la réforme, en ce qui concerne les élections européennes, le gouvernement a laissé entendre que ce serait dès début 2018, mais à ce sujet, je voulais savoir s'il est possible d'envisager un abaissement du seuil de l'attribution des sièges, c'est-à-dire que, actuellement en dessous de 5 pourcent des listes qui pourrait avoir normalement à la proportionnelle, avec une vraie proportionnelle des sièges ne peuvent pas en avoir, donc je souhaiterais savoir s'il est envisagé d'aligner ce seuil de 5 pourcent sur le seuil de 3 pourcent qui est retenue et qui me semble à mon avis très pertinent qui est retenu pour les le remboursement des dépenses électorales des euros, des élections européennes, et dernier point, on a beaucoup parlé de manière répétitive éventuelle d'un éventuel report des élections municipales pour regrouper les scrutins locaux, donc les faire passer de 2020 à 2021 il y a eu tout un tas d'annonces, un petit peu contradictoires faites par les uns et les autres, je souhaiterais donc savoir de manière. La plus claire possible et sans ambiguïté si oui ou non, le gouvernement a l'intention de reporter les élections municipales de 2020 à 2021. Merci, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Louis Masson votre 1ère question porte sur l'élection des députés, des sénateurs, effectivement, un président de la République l'a clairement énoncé au Congrès le 3 juillet dernier il. S'est engagé à proposer une réforme depuis longtemps annoncé et souhaitée par nos compatriotes tendant à réduire le nombre de parlementaires, il sera en outre introduit une part de proportionnelle au mode de scrutin pour que toutes les sensibilités soient représentées évidemment cette évolution nécessitera une évolution des circonscriptions législatives et une commission indépendante comme composée de magistrats et de personnalités qualifiées, rendra son avis sur le projet du gouvernement, vous m'interrogez sur la durée des mandats, je n'ai jamais entendu de projet dans ce sens à ce jour, ensuite vous m'interrogez sur la réforme des élections européennes, alors comme vous le savez, il a été constaté que le système en place depuis 2003, n'a ni rapprocher je dirais Les députés européens de l'heure, administré que le taux d'abstention a continué à progresser, enfin il y a eu un redécoupage, comme vous le savez, des régions et naturellement le découpage actuel à une déconnexion avec la carte des circonscriptions électorales pour les européennes, ce qui fait que, oui, on va revenir après consultation de l'ensemble dès formation politique en France,

connaissance de ce projet ou pas de ce projet de cette idée, je ne sais pas s'il y a un certain nombre d'autres personnes que vous l'ont évoqué, mais en tout cas je le note ensuite

voilà quant à la rue du cuir, du nombre d'élus locaux dont je crois, vous n'en avez pas parlé mais il n'en est pas question, bien évidemment, seule la proposition éventuelle de l'ARF de diminuer le nombre de d'élus régionaux se posent. Si Madame la Ministre, la parole est à monsieur Jean-Louis Masson pour répondre à Madame la Ministre. Madame la ministre, je prends note de de l'idée d'éventuels, de réduire le nombre des élus régionaux, sauf que c'est une très bonne idée et ça sera encore une meilleure idée si à cette occasion, mais comptez sur moi, si le débat revient au Parlement, on pouvait reposer aussi le problème du découpage complètement aberrant des régions puisque depuis qu'on a des grandes régions, pas des des pseudo grande région on a des éléments tentaculaire qui n'ont plus aucun contact avec le terrain et je crois qu'il serait certainement pertinent de solliciter l'avis des populations par le biais d'un référendum pour savoir si elle si là où il y a eu des fusions autoritaire et contre l'avis des populations concernées, on ne pourrait pas réexaminer la situation, et dernier point, la situation du projet concerne les députés et les sénateurs, j'aurais bien aimé connaître une date un échéancier de présentation au Parlement et de même, vous avez dit qu'il n'y avait pas de d'idée de réduction du des mandats dans la durée, c'est-à-dire le renouvellement des mandats, bon, c'était quand même un des éléments de la compagne du président de la République et je suis en Madame le Ministre, que vous lisiez régulièrement la presse et que vous voyez qui c'est à à dossier récurrent, on peut pas dire que personne n'en parle qu'on n'en a jamais entendu parler, ça a été au niveau des élections présidentielles et puis par la suite disons un dossier récurrent ça ça aurait pu être intéressant de voir quelle était l'intention des pouvoirs publics, notamment du gouvernement sur le sujet parce que bah disons c'est aussi je dirais dans dans la vie parlementaire intéressant de ne pas être pris au dernier moment, avoir un dossier où est en projet de réforme qui tombe du ciel, savoir exactement où on va, au cours de l'année ou des années qui viennent. Merci l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Arnaud Bazin au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la parole est à monsieur Baeza. Merci madame la présidente, la question s'adresse donc à Madame la Ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, je souhaite en effet madame la ministre vous interroger sur le projet de construction d'une caserne de gendarmerie à Beaumont-sur-Oise sur le site dit Duc ce terrain propriété de l'État car il n'existe aucun autre foncier comparable disponible et il permet de répondre à une attente légitime des gendarmes et de la population, or un avis émis par la direction générale des finances publiques en janvier de cette année, remettant en cause la faisabilité de ce projet en estimant ce bien au-delà de ce que requiert l'équilibre économique du projet telles que fixées par le loyer envisagé par votre ministère, le gouvernement précédent avait été saisi de ce dossier et le 3 mai dernier le 1er ministre en exercice avait pris bonne note de la demande d'arbitrage afin qu'une réponse soit apportée, le 6 juin dernier monsieur le ministre d'État, Gérard Collomb, répondait à madame le maire de Beaumont-sur-Oise que les services concernés seraient saisis afin d'établir un point de situation sur ce projet depuis lors, aucune information n'a été fourni, alors que ce projet est finalisé, répond bien sûr à des besoins et s'avère réalisable, pour peu que l'estimation de la valeur vénale du bien tiennent compte de l'équilibre nécessaire à l'opération par ailleurs nos réhabilitation de la caserne de gendarmerie de persan, apparaît comme une nécessité essentielle pour nos territoires, les conditions de travail de nos forces de l'ordre et un accueil digne de la population étant à l'évidence des sujets d'importance, l'état de délabrement avancé de ses locaux est inacceptable et indigne du respect que l'on doit à nos gendarmes, j'espère que c'est la seule casernes de gendarmerie de France dans laquelle on voit les racines des arbres, poussé à l'extérieur s'tendre à l'intérieur même des locaux après avoir traversé les murs madame la Ministre, ces 2 sujets étant lié pour le département du Val-d Oise je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'apporter des réponses concrètes, étant précisé que les émeutes urbaines de Beaumont-sur-Oise en 2016 ont laissé des traces, la population en conservant un souvenir très fort et très présent, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Arnaud Bazin vous m'interrogez donc sur 2 projets immobiliers concernant la gendarmerie nationale, dans le Val-d'Oise le projet de construction d'une caserne à Beaumont-sur-Oise est destiné à accueillir les locaux de services techniques et les logements des militaires servante au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de l'Isle-Adam et de l'antenne du renseignement territorial de Beaumont-sur-Oise par ailleurs, parmi les 46 logements de la future caserne parce qui bénéficierait à certains personnels de la brigade territoriale autonome de persan et aux militaires d'un peloton motorisé en cours de création cette caserne sera bâtie sur le site de l'ancien Centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, le ministre de l'Éducation nationale doit prononcer la déclaration d'inutilité de l'emprise car le bail emphytéotique signée avec l'association, qui occupait jusqu'à présent, le Centre a échu le 16 novembre dernier ce projet est désormais prise en charge par un office HLM en lien avec la direction de l'immobilier de l'État à ce stade, les partis ne sont pas encore parvenus à un accord sur les conditions de cession du site dans la valeur vénale était Sydney estimé pardon, à 1,4 1000000 d'euros par le service local des domaines l'autre projet pour partie lié au précédent consiste à réhabiliter les locaux de service de la brigade de personnes armées de 53 militaire, cette unité est installé dans un ancien commissariat de police plusieurs travaux de rénovation sont d'ores et déjà terminé en outre la reconstruction d'un abri pour les véhicules devrait s'achever au mois de janvier, tandis que les travaux de réfection des locaux vétustes commenceront au cours du 1er semestre de l'année 2018 sous l'égide de la région de gendarmerie d'Île-de-France, d'autres travaux pourraient être envisagées afin d'améliorer de manière significative l'état de la brigade, enfin une partie des militaires de la brigade de persan occupera à partir d'avril 2018 un ensemble sécurité de 33 logements situés à moins de 200 mètres des locaux de la brigade et comme je viens de l'indiquer une autre partie devra à terme être accueilli au sein de la nouvelle caserne de Beaumont-sur-Oise.

il reste un sujet qui est la réputation de la Cour de manoeuvres qui pose de sérieux problèmes mais je pense que vous avez évoqué des pistes de complément de travaux, j'espère que, on pensera à améliorer les les conditions dans la cour, parce que c'est devrait que ce sont de vraies conditions de sécurité maintenant sur l'affaire de Beaumont, le noeud du problème, c'est que le ministère de l'Intérieur, fixer un loyer et recalcul en les charges foncières qui permettent l'équipe de l'opération, on est largement en-dessous du 1000000 3 millions 4 de valeur vénale estimé il faut impérativement un arbitrage gouvernemental sur cette valeur vénale, sinon l'opération ne pourra pas se faire Val-d'Oise habitat n'ayant pas vocation à subventionner cette opération comme vous vous en conviendrez, très certainement va donc j'attire votre attention sur l'urgence de cet arbitrage, il faut qu'on Vienne à une valeur vénale du bien qui soient compatibles avec l'équilibre de l'opération, c'est le point qui reste, il est tout à fait crucial, sinon après on va dérouler toute cette opération de façon satisfaisante, tant pour les gendarmes, que pour la population que pour la ville de Beaumont-sur-Oise, merci madame la ministre.

Pemezec. Finisse mes chers collègues, le président de la République lors de la conférence des territoires, a affirmé que si on voulait que le Grand Paris fonctionne, il fallait, dans le cas de la concurrence internationale que l'on connaît, procéder à une simplification drastique des structures or 2 départements, les Yvelines et les et Les Hauts-de-Seine des élus de ces 2 départements ont anticipé les choses puisqu'ils ont décidé de fusionner, et par là même, donc de réaliser des économies d'échelle, conséquence la loi par ailleurs permet la l'article 3114 je crois 14 permet et encourage cette fusion, elle organise cette fusion et donc légalement, rien ne s'oppose à ce que ces 2 départements plusieurs puisque les 3 cinquièmes des conseils en question se sont prononcés depuis le 15 ou 16 janvier 2015, il n'y a plus d'obligation de référendum et donc il ne manque plus que le décret gouvernemental alors ma question, madame la c'est puisque ces fusions sont encouragés par l'administration et l'État puisque ces fusions procure des économies d'échelle, puisqu'on s'oriente vers une région métropole qui va donc englober à la fois des secteurs ruraux et des secteurs urbains, pourquoi le gouvernement ne signe-t-il pas ce décret est ce qu'il y aurait de d'une résistance politique quelconque, ce qui reviendrait à mettre en cause une nouvelle fois le OM décentralisation de 82 merci madame la ministre. monsieur le sénateur Philippe NZ : vous avez raison, le code général des collectivités territoriales prévoit que plusieurs départements non dans une même région peuvent fusionner par délibérations concordantes cette faculté est issu de la loi RCT de 2010 et modifié par la loi, notre de 2015, puisque non, c'est la loi de limitation des régions pardon du janvier 2005, ce qui à abroger les dispositions relatives à la consultation des électeurs de chaque département et introduit l'exigence de majorité des 3 cinquièmes de suffrages exprimés les conseils départementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont effectivement délibéré le 30 juin 2017, je veux tout d'abord souligner que le code général des collectivités territoriales précise bien que le regroupement et décidée par compte par décret en Conseil d'État et que le gouvernement n'a pas de compétences liées au recours prononcé ce regroupement, le goût, le gouvernement examinera bien sur le sujet et ce projet en fonction de considérations d'intérêt général et évidemment je ne peux pas ne pas replacer, comme vous l'fait et vous-même ce projet dans l'évolution de la métropole du du Grand Paris qui comprend dans son périmètre l'un des 2 départements concernés, en tout cas actuellement la demande des départements et des Hauts-de-Seine et des Yvelines, pourra ainsi être étudiée dès lors que les perspectives concernant la métropole du Grand Paris auront été arrêtées parce que, aujourd'hui, il y a encore des discussions une conférence territoriale spécifique qui se tiendra prochainement pour définir le cadre de travail et les perspectives permettant d'apporter des réponses institutionnelles à la hauteur des enjeux date réactivité bien sûr de ce territoire et des attentes de cohésion, de croissance et de qualité de vie de ses habitants dans cette attente, les 2 départements des Yvelines aidés Hauts-de-Seine peuvent continuer bien sûr à travailler en commun sur de nombreux sujets, comme elles le font déjà, puisqu'ils ont créé d'établissement public interdépartemental et dans les domaines d'intervention sont déjà vaste et nombreuses, mais encore une fois. Il faut bien sûr que ce projet s'inscrit dans le projet, je dirais, de la métropole Paris revue et pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin, puisqu'on ne connaît pas encore, puisqu'on est en pleine discussion voilà. Si la parole est à monsieur Pémezec pour répondre à Madame la Ministre. Merci d'un foire fois rassuré, il y a pas de blocage politique, il a juste eu une attente d'une nouvelle définition de ce que sera l'organisation territoriale de la région Île-de-France et c'est vrai qu'on souhaite tous qu'elle se simplifie cependant ça sera difficile de supprimer les départements, puis y sont inscrits dans la constitution, je le rappelle et et donc ça veut dire qu'il faudrait passer par

Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Brigitte Lherbier au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la parole est à Madame Lherbier. Même le ministre. Le domaine public est régi par de type, celui de l'inaliénabilité et celui de l'imprescriptibilité. Linda nier Bill T. du domaine public entraîne la possibilité de cession des biens du domaine public, elle suppose également que l'autorité publique propriétaire ne puisse accorder aucun droit réel une question pratique, Madame le ministre, vous voulez bien, pour lutter contre le phénomène des voitures tampons stationnant toute la journée à la même place de nombreuses communes de la métropole lilloise, ont mis en place ce qu'on appelle communément des zones bleues, ces hommes bleus viennent limiter au moyen d'un disque le stationnement des automobilistes dans la durée, elle permet ainsi au domaine public, de retrouver sa vocation initiale, c'est-à-dire un domaine de partage entre citoyens pour déroger au principe de la Zone bleue et permettra le stationnement de ses résidents ou des salariés d'entreprises situées à l'intérieur du périmètre de la Zone bleue : les mairies délivrent des cartes de résidents apposé sur les véhicules, certaines communes ont décidé de faire payer une somme modique pour délivrer ces cartes de résident en raison du principe d'inaliénabilité dont je parlais tout à l'heure d'autres communes ont choisi la gratuité, les mères m'ont demandé de clarifier leurs possibilités et de vous poser tout simplement Madame le Ministre, doit-on faire payer ses cartes de résidents, la gratuité s'oppose-t-elle vraiment au principe finale Ibn habilité du domaine public, merci Madame le ministre me répond. Merci, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Brigitte Lherbier la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique est libre car elle participe à l'exercice d'une liberté fondamentale qui est celle d'aller et venir, la liberté de stationner sur la voirie publique est un corollaire à cette liberté ainsi le stationnement est un principe libre sur la voie publique, s'il n'excède pas 7 jours consécutifs en un même point cependant, si elle ne peut être interdite de façon absolue et générale, la liberté de stationner peut faire l'objet d'une réglementation afin notamment de garantir une meilleure rotation des véhicules en stationnement, ce qui est favorable à l'environnement aux automobilistes eux-mêmes et à l'activité économique des centres villes et notamment des commerces de proximité, l'autorité investie du pouvoir de police du stationnement, maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale peut déterminer les lieux, les jours et les heures où le stationnement est réglementé

s'agissant du stationnement payant l'autorité compétente peut également édicté des tarifs différentiels entre les usagers, en raison de la particularité de leur situation, aussi est-il possible d'instaurer une tarification préférentielle gratuité ou modelé Sion pour les riverains des voies publiques, classé en zone de stationnement ayant payant pardon sans méconnaître le principe d'égalité, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil d'État l'inaliénabilité du domaine public prévue par le code général de la propriété des personnes publiques a pour conséquence d'interdire de céder une parcelle appartenant au domaine public, elle n'a pas pour effet d'interdire son occupation en outre le stationnement de véhicules sur voirie constitue une utilisation normale du domaine public routier l'instauration de la gratuité des cartes de stationnement réservé aux riverains d'une zone bleue n'est donc pas incompatibles avec l'inaliénabilité du domaine public, la collectivité en restant bien entendu propriétaire. propriétaire. Ministre, la parole est à Madame Lherbier pour une réponse à Madame la Ministre. Le ministre, je vous remercie, je ferai part aux différents maires qui m'ont posé la question de votre réponse. Merci, cher collègue. L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Agnès Canayer au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la parole est à madame canaille. Merci madame la présidente, madame la ministre mis chers collègues, ma question porte sur l'utilisation des machines à voter, c'est précisément pour lutter contre la fraude, ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin introduisit le recours aux machines à voter, à travers la loi du 10 mai 1900 conformément au code électoral, les machines à voter peuvent toujours être utilisés dans les communes de plus de 3500 habitants, elles doivent être d'un modèle agréé par le ministère de l'Intérieur, la magie a voté 2 doigts de pas être confondu avec le vote numérique ou par Internet, car elle n'est connecté L à aucun réseau, elle est une simple machine qui comptabilise les votes depuis 15 ans plusieurs communes ont fait le choix des machines à voter, Brest, Épernay et surtout Le Havre leur usage n'a jamais posé difficulté les électeurs, les élus, les agents municipaux, tous s'accordent sur la simplicité, la fiabilité et la sécurité du dispositif, malgré cela, les machines à voter suscite des oppositions souvent très doctrinal, politique rarement issus des utilisateurs, ce dispositif a d'ailleurs reçu l'assentiment à la fois du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, qui considère que le secret du vote et préservé en avril 2016, le ministère de l'Intérieur a confirmé que les fonctionnalités techniques des machines à voter, permettait de garantir la sincérité du scrutin, c'est pourquoi les villes utilisatrice souhaite pouvoir continuer à les utiliser, or depuis 2007 un moratoire interdit leur développement, les communes dotées aujourd'hui de machines à voter doivent renouveler leur parc les interdits certitude qui sur leur devenir inquiète les élus, pouvez-vous, Madame la Ministre, lever le moratoire et rassurer les élus qui utilisent aujourd'hui des machines à voter. merci, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Agnès Canayer 66 communes représentant un 1000000 d'électeurs sont à ce jour, équipés de machines à voter en 2007, à l'issue d'un travail approfondi associant le Conseil d'État, des représentants des collectivités territoriales et des usagers, le ministère de l'Intérieur et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ont décidé un moratoire ayant pour effet de figer le nombre de communes autorisées à se doter de machines à voter, comme vous venez de le rappeler les raisons qui ont justifié la mise en oeuvre de ce moratoire alors premièrement l'allongement des temps d'attente dans les bureaux équipés. je lis les conclusions qui ont été faites par les études, on coupe pour les communes et l'État entre 4000 et 6000 euros en 2007 pour l'achat d'une machine, auxquels s'ajoutent les frais d'entretien, le stockage et de formation, à une problématique de confiance de la part des citoyens devant l'impossibilité de procéder à un comptage physique des suffrages, comme l'avait relevé le Conseil constitutionnel dans ses observations sur les scrutins présidentiel et législatif de 2007, ces raisons ont été confirmés par les sénateurs, Alain Handy, Annie et Antoine Lefèvre qui ont estimé dans un rapport d'information sur le vote électronique qui est assez récent, puisqu'il est d'avril 2014, qu'il était nécessaire de proroger le moratoire contenu des risques sur le secret du scrutin et sur sa sincérité, associés à l'usage des machines à voter dans la mesure où ces dernières ne peuvent garantir ni la conformité du choix de l'électeur, ni l'absence de dysfonctionnements dans l'enregistrement des suffrages cite une phrase de leurs rapports enfin le niveau élevé de risques cyber tels que ceux qui ont récemment caractérisé les scrutins législatif et présidentiel de 2017 doit s'désormais être pris en compte dans l'appréhension des opérations de vote réalisé à l'aide de machines à voter, tenu pour une part prépondérante du père installé de l'obsolescence technique des dispositifs ainsi que du risque inhérent élevé attaché aux opérations de paramétrage des machines à voter préalables aux opérations de vote âprement par le techniques un techniques technique le gouvernement minérales Khadr applicable aux machines à voter, y compris pour ce qui concerne l'homologation à l'autorisation de nouveaux modèles de machines à voter dans le même temps, les conditions de réalisation d'un vote électronique ne reposant pas sur de tels dispositifs seront étudiés conformément au engagements du président de la République. Si Madame la ministre de la parole est à madame Agnès Canayer pour répondre à Madame la Ministre. Oui Madame il effectivement on entend les doutes et les, les, les remarques techniques qui effectivement pèsent sur les questions des machines à voter, sauf que, au quotidien, et dont l'utile l'utilisation régulière dès opérations électorales, on se rend compte qu'elles permettent quand même de favoriser le vote des personnes handicapées et qu'elles permettent aussi, donc une plus grande accessibilité qu'elle permettent aussi une plus grande rapidité dans les opérations, notamment dans celle du recensement des des votes et donc aujourd'hui, les communes qui utilisent ces machines à voter en ont pleinement satisfaction et aucun, aucun, aucune difficulté n'ont été constatés en tout cas je peux parler de mon expérience Havraises merci. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Olivier Paccaud au ministre d'État, ministre de l'Intérieur Monsieur parcours vous avez la parole. La présidente, merci Madame le Ministre, tradition oblige, les élections sénatoriales sont tous les 6 ans dans chaque département concernés par le renouvellement, l'occasion d'un vaste pèlerinage républicain tous les grands électeurs se retrouvent ensemble en un même lieu au coeur de la ville préfecture pour effectuer leur leur devoir dans l'Oise, le 24 septembre dernier les 2331 délégués sénatoriaux sont ainsi se sont ainsi rendus à Beauvais pour donc voter pour celles et ceux qui venaient du Noyonnais d'au-delà du Noyonnais d'au-delà du Valois, il aura fallu bien plus d'une heure pour venir et j'imagine que dans les départements montagnards ou dans les départements, beaucoup plus vaste, le périple vers l'urne préfectorale a pu être très long que temps passé et que dépenses que d'essence dépenser alors Madame le Ministre, à l'heure où on parle de d'économie d'énergie et de sagesse écologique ne serait-il pas plus. Rationnel et cohérent d'utiliser nos charmantes sous-préfectures de département pour s'en servir comme des bureaux de vote d'arrondissement, tout le monde y gagnerait alors si la tradition a a souvent du bon l'évolution peut parfois apporter du mieux. Si cher collègue, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Olivier Paccaud, comme vous le soulignez le code électoral désigne effectivement expressément le chef-lieu du département pour la réunion du collège électoral, en vue de l'élection des sénateurs, alors il y a 3 séries d'arguments qui motive la concentration de la réunion du collège électoral sur un lieu unique, qui peut être la préfecture. Dans mon département, c'est le tribunal. Bien, tout d'abord, une organisation du scrutin sur différents lieux seraient susceptibles de présenter un risque contentieux accrus, en effet, la réunion du collège électoral dans un lieu unique, présente l'Avantage de permettre aux préfectures chargées d'établir la liste des électeurs, de s'assurer le jour du scrutin, de l'identité de l'ensemble des électeurs et de vérifier à l'appui d'un document unique que les demandes de remplacement ont été correctement formalisé et remplissent les conditions fixées par le code électoral, je rappelle que c'est la seule élection en France qui soit obligatoire en outre une démultiplication des lieux de vote pourrait engendrer plusieurs difficultés pratiques, elle pourrait compliquer l'exercice par le bureau du collège électoral de ses missions en effet les attributions conférées à ce bureau qui remplit également le rôle de bureaux de la 1ère section rend nécessaire une proximité physique avec les autres sections le jour du scrutin, seul le président du bureau du collège électoral est habilité à statuer sur les difficultés et les contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, toutes sections confondues, cette concentration permet également aux représentants de lys d'accomplir leur mission de contrôle des opérations de vote dans l'ensemble des sections de vote enfin cette concertation sur un site unique est un moyen de garantir au mieux l'accessibilité à tous les électeurs des résultats proclamés par le bureau du collège électoral pour l'ensemble du scrutin, compte tenu notamment du court délai 4 qui sépare les 2 tours dans le cadre du scrutin majoritaire à 2 tours, enfin il ne faut pas aussi dit mais, Monsieur le Sénateur, l'intérêt au fond politique, de la réunion du collège électoral, on allie unique dans la mesure où cette dernière constitue une opportunité d'échanges entre élus s'ouvrant apprécié de ces derniers, j'ai bien entendu les arguments écologiques que vous avez soulevé, mais pour toutes ces raisons, le gouvernement n'est pas favorable à l'organisation de modalités d'élection différentes pour les sénatoriales. à parole est à monsieur Olivier Paccaud pour répondre à Madame la Ministre. Merci à un minutes pour votre réponse, qui n'a pas du tout convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, il y avait des arguments écologiques, il avait des arguments économiques et en matière d'économie, vous nous donnez des leçons vous donnez sont constamment aux collectivités le fait de rapprocher les grands électeurs de leur bureau de vote qui permettrait de réelles économies alors certes pas c'est pas énorme, mais alors que vous ne cessez d'encourager d'exhorter les collectivités, économie, il serait bon de montrer l'exemple, nous sommes sous la IIIe République et l'égalité devant le scrutin, nous ne sommes vraiment pas du tout mise à Bâle par le fait d'avoir, dans l'Oise, il y a 4 sous-préfectures qui est 4 bureaux de vote, voilà, alors j'ai bien compris, vous vouliez pas bougé ben écoutez, nous en sommes à la 5ème République mais peut-être que la 6ème République fera un petit peu plus intelligente. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle à questions orales de Monsieur Claude rénal au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la parole est à monsieur rénale. Oui merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues permettez-moi de commencer cette question par quelques chiffres en 2016, 60 pourcent des enfants sont nés hors mariage en France et toujours en 2000 16 heures 44 pourcent des mariages finissent par un divorce la parentalité ne s'exerce non plus que minoritairement dans le cadre d'un mariage s'il appartient au juge civil d'encadrer les questions de garde et de résidence d'autorité de pensions ou de logements entre les parents, il ressort que l'administration aussi un rôle à jouer en ce qui concerne la délivrance de papiers d'identité aux enfants, en effet, les services municipaux chargés de la délivrance Titre non juridiquement pas l'obligation de rechercher si le parent demandeurs et qui tue l'air de l'autorité parentale ou que l'adresse déclarés et celle de la résidence principale de l'enfant, aucun des documents à fournir ne contient cette information pourtant importante au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, tout au plus, nos textes prévoient qu'il appartient aux parents, titulaire de l'autorité parentale, d'en faire la demande, mais l'absence de contrôle de l'effectivité de la détention de cette autorité rendent bien illusoires cette protection purement formelle dans l'hypothèse de parents séparés ce défaut de contrôle des informations se doublent d'une absence d'information de l'autre parent qui n'apprend alors que fortuitement lorsque lui-même en fait la demande de l'existence des autres papiers d'identité s'était a, de fait, entraîne une situation quelquefois d'anxiété chez le parrain de bonne foi, d'autant plus grande que cette pièce d'identité, bien plus que les autres permet un éloignement non consenti de novembre d'un enfant français de son sol d'origine sans possibilité pour l'autre parent de s'y opposer, problème, un autre sur la situation de l'enfant vis-à-vis de l'administration, cette dernière ne reconnaissant que la validité de la dernière domiciliation l'administration faisant alors porter la charge de la preuve, l'existence d'une fraude non pas sur l'émetteur de la demande litigieuses, mais sur celui qui la qui la contestent, en outre, le parent indélicats peut aussi lors de sa demande, déclaré le titre précédent lui ce qui peut entraîner des situations juridiquement 4ème pour le port de bonne foi, enfin, au-delà de la difficulté de se qui situation préparant séparer mon interrogation vise aussi à alerter aussi d'une possible responsabilité de l'administration en cas de départ non consenti de l'enfant du territoire national par exemple, l'on sait que ces questions peuvent prendre relief particulier dans le contexte actuel, aussi je souhaiterais connaître madame la Ministre, la position de votre gouvernement, face à ce problème qui peut concerner éventuellement des millions de nos concitoyens. monsieur Reina, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Claude rénal, vous m'interrogez sur la réglementation applicable en matière de délivrance de passeports pour les enfants mineurs dont les parents sont séparés et dont le consentement d'un des 2 détenteurs de l'autre hériter. Parental n'ait pas exprimé en effet l'article 372 tiré 2 du Code civil prévoit qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents et réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait, seul un acte usuel de l'autorité parentale, relativement à la personne de l'enfant, la demande de titre d'identité et de voyages pour un enfant mineur, est considéré comme un acte usuel de l'autorité parentale, en outre, la séparation des parents ne modifie pas, sauf disposition contraire du juge le partage de l'autorité parentale ainsi la demande de titres pour un enfant peut être déposée par l'un des parents, sans qu'il soit nécessaire de demander effectivement l'accord de l'autre parent le formulaire de demande de titre de voyage impose aux demandeurs par la position de sa signature de certifier l'exactitude des mentions et déclarations qu'il y a porté toute force de déclaration et est passible d'une peine d'emprisonnement et d'amendes prévues par le code pénal, ainsi il n'a appartient pas aux mairies, vous l'avez dit lui-même, vous-même, pardon, chargé du recueil de demande de passeport de solliciter l'accord de l'autre parent, ni aux services instructeurs de rejeter une demande de passeport, déposée par un seul parent si aucune opposition en la matière n'a été préalablement manifesté en cas de conflit entre les parents, liée au partage de l'autorité parlons ou en cas de crainte de l'un des parents de voir un enfant emmené à l'étranger sans son accord, il lui appartient de saisir le juge aux affaires ne familial qui prononcera le cas échéant, une mesure d'interdiction du sortie de territoire dans l'attente de la décision du juge le Parenti craint l'enlèvement de son enfant, peu sollicité auprès de la préfecture, une mesure d'opposition à la sortie du territoire de l'enfant mineur, il s'agit d'une mesure prise à titre conservatoire, qui a pour objectif de permettre aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant, dans l'attente d'obtenir, en référé, une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire, voilà l'état du droit monsieur rénale, mais c'est vrai que c'est une vraie question que vous posez. Madame la Ministre Monsieur rénal pour répondre à Madame la Ministre. D'abord pour la remercier de sa réponse et si elle ne permet de le remercier de sa petite dernière phrase parce que je crois que l'état du droit effectivement hé hé bien pauvre par rapport à la problématique est telle qu'elle se présente actuellement à la fois en quantité et à la fois par rapport aux sujets que nous connaissons quelquefois bien dramatique et sur lesquels faire référence au juge des enfants, préventivement, etc, hé, hé, hé, hé bien complexe et ne résout pas vraiment le sujet je pense que ce qu'il faudra regarder peut-être à l'avenir, c'est si c'est par le truchement d'un texte de loi, je ne sais pas, ou si c'est par un règlement ou un décret que le voir dès qu'une information des mairies, que les choses devaient être traitées de manière me semble-t-il, plus solide, en tout cas j'appelle à ce qui est une réflexion du du ministère sur ce sujet et que l'on vieillit bien me dire s'il y a de quoi : nécessité d'avancer par une proposition de loi ou d'autres solutions finalement technique permet de répondre à la question posée, je vous remercie. Si chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Michel à 9 et à la ministre de la culture, vous avez la parole chers collègues. Merci madame la présidente, mesdames les ministres, chers collègues, je souhaitais effectivement interroger Madame la ministre de la culture sur le fonctionnement de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, qui est un institution importante dans notre pays puisqu'elle défend les droits de près de 160000 membres adhérents de cette institution elle perçoit pour cela, j'ai tout à fait conséquents en l'occurrence les droits de diffusion de musique pour un montant légèrement inférieur à 1 milliard d'euros, c'est donc une société qui est importante et puis nous avons à côté de cela sur notre territoire un certain nombre d'organisateurs de manifestations diverses, souvent ce sont des associations qui organisent différentes animations telles que des balles, tels que des repas et puis tout autre manifestation et donc ces manifestations peuvent avoir recours à à à des prestations de musique

c'est de la musique qui existe déjà depuis très longtemps et qui est donc joué dans différentes animations culturelles territoriales et donc c'est les associations sont souvent sollicités par la Sacem pour payer des droits, alors quand il y a des recettes qui sont conséquentes, ça va bien et puis quand il y a peu de recettes, c'est difficile pour ces associations, hé bien souvent, le doute est mis sur le fait qu'elles doivent payer les droits pour ce qui concerne le fait de pratiquer la musique traditionnelle populaire régionale et donc je souhaitais interroger le gouvernement à ce sujet, Madame la Ministre, et savoir comment on pouvait interpréter cela et comment c'est organisateurs pouvaient éventuellement être dispensé de payer les droits, s'il s'agit de morceaux qui sont déjà dans le Patrimoine général depuis très longtemps.

le sénateur Canuet, Madame la sénatrice, vous interrogez le gouvernement au sujet du versement d'une rémunération pour l'exécution des musiques traditionnelles bretonnes, tombé dans le domaine public, à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, comme vous le savez, le code de la propriété intellectuelle, précise que la durée de protection d'une oeuvre musicale et de 70 ans après la mort, le décès de son compositeur à l'expiration de ce délai, le vrai peut être exploité librement peut être exploité librement sous réserve du droit moral de l'auteur, bien sûr, et gratuitement, la Sacem n'a donc pas vocation à percevoir de rémunération pour la diffusion d'une oeuvre musicale dans l'du même public, sauf dans l'hypothèse où cette eau ferait l'objet d'arrangements ou d'adaptation dans le cas de l'association que vous relevez les morceaux exécutés n'ont fait l'objet d'aucune adaptation susceptibles de donner naissance à des droits d'auteur et donc, comme le prévoit la législation en vigueur pour toute manifestation musicale sachez donc, Monsieur le Sénateur qu'après examen du programme des Oeuvres interprétées par ce groupe d'accordéonistes dont vous faites mention le dossier a été clos par la Sacem et n'a donné lieu à aucune suite administrative aux facturations à titre de droits d'auteur. Merci madame la Ministre, la parole est à monsieur Canivet pour répondre à Madame la Ministre. Merci madame la Ministre pour votre réponse, effectivement, il était important de clarifier les choses et en particulier de bien mettre en évidence que lorsqu'il s'agit de 2000 morceaux de musique traditionnelle ancienne et bien qu'il n'y a pas de droits à payer dès lors qu'effectivement il n'y a pas eu d'arrangements particuliers donc je remercie tout à fait pour votre réponse qu'on administre. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Catherine Dumas à la ministre de la culture, la parole est à Madame Dumas. Merci madame la présidente, madame la ministre, comme tous mes collègues sénateurs de membres de la commission culture, éducation et communication, j'ai été mise en copie de 2 alertes qui vous ont été adressées par un représentant du personnel de l'Opéra de Paris, le 27 septembre le 17 octobre s'agissant de dégradations qui seraient dans la salle et les loges du Palais Garnier, alors s'il est avéré, le reportage photo qui était joint d'ailleurs assez alerte est assez édifiant avec des boiseries détérioré des tapis usés des fauteuils dégradé tapisseries de l'abri etc l'Opéra de Paris bien sûr est un monument historique classé en 1923 c'est un des édifices structurant de la capitale, mais c'est aussi une des vitrines du Patrimoine français, alors que le président de la République a fait du Patrimoine, un axe prioritaire de son action culturelle, vous l'avez d'ailleurs, Madame la Ministre rappeler hier dans cet hémicycle, je suggère qu'une inspection soit diligentée par votre ministère afin que des explications soient apportées sur la préservation de cette salle de renommée mondiale, le cas échéant, bien sûr, je souhaiterai connaître à travers un état des lieux, le plan de mesures évidemment de travaux de réfection qui mettra à contribution les savoir-faire des artisans d'art français. Si Madame Dumas, la parole est à madame la ministre de la Culture Madame Françoise Nyssen. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, comme nombre de vos collègues parlementaires vous interroger le gouvernement sur la situation de l'Opéra Garnier je voudrais d'abord vous dire alors que comme vous le disiez votre assemblée a voté et adopté hier les crédits budgétaires de notre ministère, je tiens à rappeler que les investissements réalisés à l'Opéra national de Paris, c'est-à-dire le Palais Garnier, l'opéra Bastille, l'école de danse et les Ateliers Berthier qui accueille près de 1,6 millions de spectateurs et visiteurs chaque année et plus de 1500 salariés chaque jour sont de lors de 10 à 12 millions d'euros pour 2018 la subvention d'investissement il concourt à quoi s'ajoutent les ressources propres de l'établissement, il y a la capacité d'autofinancement générée par ce chaque année par son activité, ses 6 millions d'euros environ environ la mise à contribution éventuelle en complément du fonds de roulement et les ressources de mécénat affectés à certains opération de travaux concernant plus particulièrement la salle du Palais Garnier un programme de rénovation effectivement comprenant la restauration de tissus délogent des fauteuils recréer de l'éclairage, le déplacement des projecteurs et aussi de la zone publique a été établi en août 2014 et mises en oeuvre depuis le programme de rénovation de la salle va se poursuivent pour un coût total d'environ 2,5 millions d'euros, ces 4 prochaines années, et les rénovations de la galerie et celle de la Rotonde du glacier pourrait-elle faire l'objet d'un financement par voie de mécénat les opérations d'investissement de l'Opéra national de Paris font l'objet d'un plan pluriannuel d'investissement examiner régulièrement par les ministères de la culture et du budget, et soyez assurés que mes services assurent un suivi attentif et accompagne d'établissement dans ces rénovations d'ampleur et dans l'importante transition qui représente de transfert de la maîtrise d'ouvrage du bâtiment du palais Garnier. Merci madame la Ministre, la parole est à Madame Dumas pour répondre à Madame la ministre. Merci madame la présidente, madame la ministre, tout d'abord je voudrais vous remercier d'abord de vous être déplacé personnellement au Sénat pour répondre à ces 2 questions qui sont de votre domaine vous remercie également de votre réponse, vous dire qu'en tant qu'élu de Paris, bien bien sûr, je suis également très sensible à ce que vous avez répondu à ce plan de rénovation et qui serait évidemment particulièrement attentive à la suite, qu'il sera donné. Merci, cher collègue, j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations ont été publiés ces candidatures seront ratifiés si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Je vais suspendre la séance 7 sera reprise à 14 heures pour la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, la séance est suspendue.